Nous poursuivons l'examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les États généraux de l'alimentation, nous nous attendions à un budget généreux de l'agriculture. Or, ce que nous constatons, c'est une mise au régime sec, peut être en écho aux épisodes de sécheresse que les agriculteurs ont eu à subir cet été. À le lire, monsieur le ministre, j'ai l'impression d'être déjà en pleine période de carême En termes plus économiques, c'est à un budget sans vitalité macroéconomique et aux impacts microéconomiques tout à fait inacceptables que nous sommes confrontés. Lors de la discussion de votre budget à l'Assemblée nationale, vous avez indiqué que « ce qui compte, ce n'est pas sa masse budgétaire ». Permettez-moi de m'étonner, car nous savons bien que la masse budgétaire, cela compte pour un budget dont la vocation primordiale est d'accompagner les efforts de nos agriculteurs, de leur permettre de vivre de leur activité et d'offrir aux Français toutes assurances de pouvoir consommer des produits sains. N'oublions pas, monsieur le ministre, que la moitié des agriculteurs de ce pays dispose d'un revenu annuel avant impôt de 14 000 euros, et qu'entre 15 % et 25 % des agriculteurs n'ont tout simplement pas de revenu. Faut-il aussi rappeler ici le désespoir de bon nombre d'exploitants ? Faut-il rappeler encore le nombre de suicides constatés dans le secteur agricole ? La France perd, année après année, des exploitations, et l'emploi agricole a chuté de près de 60 000 postes depuis 2010. La valeur ajoutée agricole est volatile, mais c'est surtout sa croissance qui s'est de longue date volatilisée. La situation agricole de ce pays appelle un redressement ; la situation de nos agriculteurs mérite davantage de respect et de considération. Avec des crédits inertes, le budget que vous défendez n'est pas à la hauteur de ce défi économique. Il n'est pas davantage au rendez-vous des deux ambitions majeures que devrait porter ce pour la vitalité des territoires ruraux, et une agriculture en transition vers un horizon agroécologique. Monsieur le ministre, sans moyens réels, que devient l'objectif de convertir 15 % de la surface agricole française au bio dès 2022,

? Ne vous appuyez pas sur la hausse des crédits de l'ICHN, car vous savez bien qu'elle est financée par les agriculteurs et qu'au niveau de chaque exploitation elle n'apportera pas un centime de plus. Ce budget sans élan est également inacceptable d'un point de vue microéconomique. Une dotation pour dépenses imprévues a été intégrée au budget pour 2018. Comme c'était à craindre, elle n'a couvert que des dépenses prévisibles, celles nécessaires pour couvrir les corrections financières arrêtées par la Commission européenne pour sanctionner des défaillances de gestion des aides par votre ministère. Il reste un reliquat. Comptez-vous l'employer pour compenser les aléas de production dus à la sécheresse ou bien pour compléter des lignes budgétaires insuffisamment dotées ? Vous entendez réduire d'un tiers cette dotation, en vous fondant sur la consommation des crédits de 2018, c'est-à-dire sur une dette d'apurement de l'ordre de celle réglée en cours d'année. Compte tenu des risques pendants, cela paraît bien imprudent, cela signifie que vous ne disposez dans le budget initial de 2019 d'aucune marge pour soutenir les exploitants. Cela n'est pas acceptable Et la déduction pour épargne de précaution ne changera rien à l'affaire pour la plupart des agriculteurs. Dans le sombre panorama de l'emploi agricole, le seul type d'emploi qui conserve un peu de dynamisme, c'est l'emploi saisonnier. Eh bien, voilà que vous le pénalisez, monsieur le ministre ! La réforme

Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à nous annoncer un plein retour au dispositif en vigueur ? J'en finirai avec quelques mots sur le CASDAR. Nous souhaitons ici que la recherche soit pleinement intégrée à notre politique agricole. Il serait au demeurant souhaitable que l'INRA devienne un opérateur de la mission. Nous sommes inquiets de voir le CAS accumuler des moyens qu'il n'est pas en mesure de dépenser, selon les critères admis d'évaluation scientifique. Nous pressentons que, bientôt, le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations qui doit alimenter l'innovation agricole sera détourné de son objet pour des usages sans aucun lien avec l'agriculture.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous savez l'intérêt porté par cette assemblée à l'agriculture et la place qu'elle occupe dans la vie des territoires. Nous sommes convaincus que cette activité est stratégique et qu'elle constitue une garantie de non-dépendance dans un monde instable et balayé d'incertitudes. En outre, nous percevons bien à quel point nos concitoyens sont plus que jamais vigilants et réactifs s'agissant des conditions de la production agricole, ainsi que de la qualité de l'alimentation. Par ailleurs, nous savons que nous vivons une période particulière. Le réchauffement climatique suppose de se préparer- il n'est que temps ! -aux aléas qui devraient s'accentuer et affecter l'agriculture, comme il faut faire face aux nouveaux risques sanitaires qui se manifestent à épisodes rapprochés désormais peuvent surgir à chaque instant dans un monde rétréci par la mobilité. Chacun connaît les conséquences de la fièvre catarrhale ovine, du virus H5N1, qui en est d'ailleurs à la quatrième ou cinquième génération désormais, sur l'économie des filières. Aujourd'hui, c'est la peste porcine présente en Pologne qui fait peser un risque substantiel sur cette production. dit pour rappeler, monsieur le ministre, que le budget doit répondre à deux sujétions : celle du court et du moyen terme, bien entendu, mais aussi celle de l'avenir, Le sentiment que j'éprouve est que, pour une part importante, le budget poursuit sur sa trajectoire antérieure pour une grande part des dépenses qu'il prévoit, et ce dans l'attente de deux éléments déterminants la nouvelle politique agricole commune et les conséquences du Brexit, sans doute difficiles à évaluer complètement à ce stade. Du point de vue du contexte économique, le ministre de l'agriculture de 2018 se et c'est heureux, dans une situation plus apaisée que son prédécesseur l'an passé, la conjoncture agricole s'étant améliorée, même si elle demeure atone. Par ailleurs, vous bénéficiez des efforts accomplis antérieurement afin d'améliorer le fonctionnement de la chaîne de paiements agricoles, ce qui devrait nous épargner de lourdes corrections financières européennes. Ces événements demeurant néanmoins aléatoires, tout relâchement des efforts de provisionnement des risques et de modernisation du cadre de gestion doit être exclu. On doit à cet égard regretter la réduction de la dotation pour imprévus, ainsi que les variations autour du financement de la nécessaire modernisation des systèmes de l'Agence de services et de paiement. paiement. L'avenir de l'agriculture mérite incontestablement mieux qu'un simple budget de reconduction, d'autant, monsieur le ministre, que nous devons, notamment, nous engager résolument vers une production plus diversifiée, biologique en particulier, qu'il ne s'agit pas, ainsi que vous l'avez plusieurs fois indiqué, d'opposer à l'agriculture conventionnelle, elle-même en voie de redéfinition. Vous évoquez, monsieur le ministre, l'allégement des cotisations sociales, qui se traduira par un renforcement des transferts vers la production agricole. Localement nous sommes surtout interpellés sur l'intérêt de conserver le régime TO-DE, qui concernerait 70 000 exploitations. il n'y a pas forcément adéquation entre l'emploi salarié en général, qui est loin de concerner toutes les exploitations, et l'emploi propre à certaines productions et l'emploi propre à certaines productions saisonnières ; je pense en particulier à la filière légumière, mais l'on pourrait tout autant citer l'arboriculture, que vous connaissez particulièrement bien, voire la production de sapins de Noël, comme l'a rappelé un collègue de la Nièvre. Nièvre. La filière bois, quant à elle, demeure très déficitaire au titre du commerce extérieur, alors que la forêt française est la plus vaste d'Europe. J'ouvre une parenthèse, afin de vous rappeler le rapport parlementaire produit par le Sénat, à ce jour resté sans écho. Qu'envisagez-vous de proposer afin de relocaliser la transformation de la ressource, donc la valeur ajoutée ? Le Gouvernement a signé récemment un nouveau contrat de filière avec les professionnels du bois. Quelle stratégie induit-il, monsieur le ministre ?

La qualité sanitaire de nos productions et de l'alimentation sera en permanence un sujet de préoccupation, comme tout ce qui concerne la santé publique. Le programme 206 finance une partie des dépenses correspondantes. Or il demeure à peu près inchangé, une fois pris en compte l'éventuel dénouement particulièrement laborieux du contentieux des vétérinaires sanitaires. Est-il opportun de maintenir simplement cette dépense quand tout, autour de nous, invite au contraire à l'accentuer ? 40 emplois sont créés pour anticiper les effets du Brexit et les détournements de trafic qu'il occasionnera possiblement, et même certainement. C'est assurément trop peu compte tenu de besoins de contrôle dont, je l'accorde volontiers, on ne sait quand ils se matérialiseront complètement. Nous sommes en permanence confrontés à l'irruption et la propagation de crises sanitaires toujours lourdes de conséquences économiques et financières pour les producteurs. Ni l'influenza aviaire, dont de nouvelles souches existent de par le monde,

une meilleure organisation pourrait permettre des gains d'efficacité. Sur ce sujet encore, nous avions proposé, dans un rapport de la commission des finances du Sénat, de repenser et réorganiser notre infrastructure de maîtrise du risque. et du travail, est quelque peu renforcée. La perspective du Brexit pourrait ne pas y être pour rien, puisque 40 % des autorisations de mise sur le marché, les AMM, des médicaments vétérinaires seraient aujourd'hui accordées au Royaume-Uni. Or il existe pour le moins quelques sérieux problèmes du fait de la concurrence pouvant exister entre les intervenants participant à la délivrance des AMM. Cet aspect du rôle de l'ANSES a été beaucoup développé, malgré l'écart entre les coûts qu'il entraîne pour l'agence et les retours financiers qu'elle perçoit. Je relève que ce déficit serait de nature à peser sur les autres activités de l'ANSES au service de la recherche et des opérations courantes d'identification de nouveaux risques sanitaires. Au-delà, alors que nos compatriotes s'inquiètent des effets des produits, phytopharmaceutiques notamment, il faut s'interroger sur les conséquences de cette situation concurrentielle entre agences sanitaires. ministre, il convient que nous soyons attentifs, dès aujourd'hui, à l'impérieux devoir de recherche, pour prévenir les conséquences des changements climatiques, par la mise au point des semences plus résistantes et par l'accès à des techniques de production plus adaptées aux nouvelles conditions. En un mot, il faut que nous soyons pleinement préparés à ce bouleversement, pour maintenir notre économie agricole.

monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année 2019 est l'année de toutes les incertitudes pour l'agriculture. Le moment était venu d'envoyer un vrai signal à destination des agriculteurs. Il l'a été, mais, malheureusement, ce n'est pas le bon. C'est donc au moment où le budget de la PAC est sur le point de diminuer de 15 % en euros constants que le budget de la mission recule de plus de 200 millions d'euros, soit 10 % à périmètre constant. C'est donc au moment où les aléas n'ont jamais été si forts pour l'agriculture française, vous le savez, monsieur le ministre, que la réserve pour aléas, créée l'année dernière, voit ses crédits amputés d'un tiers. C'est donc au moment où la concurrence n'a jamais été aussi forte sur nos productions que l'un des dispositifs les plus efficaces en faveur de la compétitivité de certaines filières, à savoir le TO-DE, est supprimé. Tous ces paradoxes ne font que révéler l'ambiguïté de la politique agricole gouvernementale. Il faut rétablir la vérité La vérité, c'est que la réserve de crise du budget agriculture n'en est pas une. Elle ne sert qu'à financer des apurements communautaires. Aucun euro n'a été déboursé cette année contre des aléas agricoles ; pourtant, monsieur le ministre, si vous les interrogez, Cette réserve ne revient nullement aux agriculteurs en cas de calamités. Elle n'est qu'une épargne que l'État conserve pour couvrir chaque année les dépenses induites par les erreurs de son administration. La vérité, c'est que la loi ÉGALIM ne peut réellement inverser le rapport de forces entre les producteurs et leurs acheteurs que si les contrôles du bon respect des contrats sont appliqués. Or ce PLF réduit les effectifs des deux instances chargées de ces contrôles : la DGCCRF et FranceAgriMer C'est à se demander, monsieur le ministre, si le Gouvernement ne doute pas de l'efficacité de sa propre loi ! La vérité, c'est qu'il n'est pas envisageable d'avaliser cette réduction du budget de l'agriculture, alors même que l'agriculture en a tellement besoin. C'est en tout cas le point de vue de la commission des affaires économiques et le mien. En conclusion, monsieur le ministre, je vous demande de cesser ce jeu de massacre, qui consiste à stigmatiser sans cesse notre agriculture.

et sommes de plus en plus tributaires de l'importation de produits étrangers qui ne respectent ni nos normes ni nos façons de produire. Monsieur le ministre, réagissez, et réagissez très vite

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur la sécurité sanitaire. La France dispose de l'un des meilleurs systèmes au monde. C'est ce que rappelle un récent classement international. Même si le risque zéro n'existe pas, et c'est tout le problème, il faut en être fier. Ce n'est pas pour autant que la France doit se reposer sur ses lauriers. Les défis sanitaires auxquels elle va devoir faire face sont nombreux, comme en témoigne le risque d'épidémie de peste porcine auquel la France est désormais exposée. Or le budget du programme « Sécurité et qualité sanitaires » affiche un recul, certes comptable, mais un recul tout de même. Parmi les principaux problèmes posés à notre sécurité sanitaire, le Sénat n'a de cesse de dénoncer les importations de denrées alimentaires de pays tiers ne respectant pas les normes européennes. Les résultats des contrôles aux importations sur ces produits sont en effet très préoccupants. On peut estimer aujourd'hui qu'au moins un produit importé de pays tiers sur dix ne respecte pas les normes sanitaires et phytosanitaires européennes. Il est parfois de plus de 25 %. Rien que pour les produits issus de l'agriculture biologique, il est, par exemple, de 17 %. Je vous laisse y réfléchir, Et ces chiffres ne prennent pas en compte le taux de non-conformité des importations venant de pays de l'Union européenne, plus difficile à mesurer, et sans doute encore plus élevé. Cette situation est intenable ! D'une part, elle pose d'immenses problèmes sanitaires, car ces importations nuisent à une bonne protection des consommateurs. D'autre part, ces importations constituent une concurrence déloyale massive pour nos agriculteurs français. Comment peut-on leur demander d'augmenter leurs standards de production tout en favorisant l'importation de produits ne les respectant pas ? Le seul moyen de lutter contre ce phénomène, c'est d'accentuer les contrôles et de renvoyer une fois pour toutes tous les produits non conformes pour faire comprendre aux autres pays que la France est inflexible. Comment voulez-vous assurer un contrôle efficace quand l'État dépense moins de 10 millions d'euros par an pour contrôler l'ensemble des denrées alimentaires importées ?

Trois tirages du Loto pour la sécurité sanitaire des Français et la compétitivité de notre agriculture, cela ne paraît vraiment pas cher payé. Depuis la loi ÉGALIM, l'autorité administrative doit prendre toutes les mesures de nature à faire respecter le principe d'interdiction à la vente de produits non autorisés dans l'Union européenne. Il est temps, monsieur le ministre, de prendre les mesures exigées par la situation et, surtout, de répondre aux obligations fixées par la loi. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tant que j'aurai de la voix, je dirai et redirai ce chiffre effroyable, qui a déjà été évoqué : un agriculteur se suicide tous les deux jours ! Pour quelle autre profession accepterait-on ce tragique constat ? Monsieur le ministre, vous l'avez dit vous-même sur ces travées, les lois agricoles se succèdent, mais rien n'y fait. Ce malaise paysan reflète le malaise de notre société, car les enjeux que l'agriculture englobe sont universels indépendance alimentaire, qualité alimentaire, santé publique, emplois non délocalisables, attentes sociétales, aménagement du territoire, lutte contre les incendies. Vous avez affirmé une ambition pour la politique agricole. Pour vous avoir côtoyé de près dans vos combats dans nos rangs au Sénat, je crois en votre sincérité et en votre connaissance du terrain. Pour autant, vous le savez, ce n'est pas vous seul qui allez décider. Pour concrétiser des ambitions, il faut s'en donner les moyens, et ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux de l'agriculture française. Parlons méthode, tout d'abord. Votre prédécesseur avait mis en place les États généraux de l'alimentation. J'avais salué et même participé à ces ateliers, qui consistaient à placer autour d'une même table tous les acteurs de la chaîne. L'intention s'est arrêtée en cours de route : la loi ÉGALIM a permis quelques avancées, mais elle a provoqué les inquiétudes des filières et des organisations syndicales. Face à la guerre des prix de la grande distribution, la recherche d'un prix juste pour le producteur n'a rencontré aucune solution. La suppression annoncée de l'allégement des charges pour les TO-DE, maintenu, mais à la baisse, jusqu'en 2020, malgré une volonté forte du Sénat de pérenniser cette mesure, nous entraînera forcément à une perte de compétitivité.

La Chine, le Brésil, les États-Unis, qui ont bien compris les enjeux d'une politique agricole engagée et soutenue, ont augmenté leur budget pour soutenir leurs filières. Dans un contexte mondialisé et de libre-échange, où notre compétitivité se heurte à des iniquités tout aussi sociales que normatives, nous avons de grands doutes sur l'avenir de notre politique agricole commune.

rendez-vous dans un an, mais je pense que, malheureusement, il n'y aura eu aucune redistribution de la valeur. Les paysans, une fois de plus, en subiront les conséquences et resteront dans le désespoir. Mes Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

le mercredi 18 avril 2018 au matin, alors que j'étais en commission des affaires étrangères, j'ai reçu un message qui m'a bouleversé : mon neveu Jean-Louis, agriculteur, venait d'être retrouvé mort au volant de son tracteur. En prenant la parole aujourd'hui, je souhaite lui rendre hommage, ainsi qu'au monde agricole, qui travaille par amour de la terre au prix de nombreux sacrifices et pour de faibles rémunérations. Notre monde est aujourd'hui confronté à des enjeux capitaux : changement climatique, explosion démographique, épuisement des énergies fossiles, vieillissement et dépendance, inégalités croissantes, déséquilibres socio-économiques, perte de biodiversité. Tous ces défis sont complexes, car ils sont interdépendants. Ils nécessitent l'alliance de nombreux acteurs, s'inscrivent dans le long terme et ne s'accommodent pas de réponses simplistes. Une chose est sûre : l'agriculture, que ce soit à l'échelon national ou au niveau européen, a un rôle crucial à jouer. L'agriculture française présente un bilan de santé contrasté. Si la France compte des champions agro-industriels, des entreprises intermédiaires innovantes très compétitives sur des marchés mondialisés, plusieurs signaux d'alerte montrent que le secteur vit des mutations profondes et souvent douloureuses. De nombreuses exploitations sont aujourd'hui en détresse, et un agriculteur sur quatre en France vit sous le seuil de pauvreté. Les raisons de cette paupérisation sont bien connues : elles tiennent à la fois à la dérégulation des marchés agricoles et, surtout, à la très inégale répartition de la valeur dans les filières agricoles et alimentaires. La profession d'agriculteur est le deuxième métier le plus dangereux au monde, avec des conditions de travail difficiles, un isolement fort, des accidents de travail bien trop nombreux. Nous avons, en tant qu'acteurs publics, une responsabilité à assumer face à ce triste constat. C'est la catégorie

Eu égard à l'enjeu humain, ce projet de budget 2019 n'est pas assez ambitieux : relativement stable, il s'inscrit dans la continuité d'une politique menée depuis des années, avec la reconduction de la plupart des dispositifs. Il prend trop peu en compte les grands défis auxquels est confronté ce secteur. Il faut absolument adopter un nouveau regard sur l'agriculture française, changer de paradigme en matière de politiques publiques pour favoriser et mieux prendre en compte la diversité des agriculteurs et des agricultures. Il convient également de la sécuriser, de la valoriser et de la rendre plus attractive, pour qu'elle soit durable, équitable et performante. La sécuriser, car 2019 sera sans conteste une année charnière pour l'agriculture, qui fera face à de nombreuses incertitudes, incertitudes, avec notamment la gestion du Brexit, la réduction de 15 % des crédits de la PAC, et une concurrence toujours plus forte, souvent trop déloyale. La réforme de la fiscalité agricole reste trop frileuse pour sécuriser le secteur agricole. Nous pouvons saluer le dispositif unique de déduction reposant sur la constitution d'une épargne de précaution. Cela permettra d'aider nos agriculteurs à faire face aux aléas de plus en plus fréquents grâce à des outils fiscaux leur permettant d'améliorer leur résilience et leur compétitivité, tout en leur assurant des revenus stables. Nous approuvons aussi le maintien du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques sur le secteur non routier pour l'agriculture. nous ne pouvons, en aucun cas, soutenir la suppression du dispositif d'exonération des charges pour les travailleurs saisonniers. Je salue d'ailleurs la position du Sénat, qui a défendu le maintien en sa forme actuelle au-delà de 2021, et la dernière position de l'Assemblée nationale, qui semble tendre vers un compromis acceptable. Nous regrettons également la diminution des crédits prévus pour la réserve de crise et considérons qu'il serait souhaitable d'augmenter davantage les fonds à destination des zones à handicap naturel. Nous souhaitons que soient valorisées nos filières agricoles en soutenant davantage l'enseignement agricole. Le budget restera stable en 2019. Il faut diversifier leurs activités, promouvoir les filières innovantes. Il s'agit de relever le défi et d'anticiper les métiers de demain. Cette valorisation passe également par une meilleure communication sur la sécurité alimentaire des productions agricoles françaises : les règles sanitaires appliquées sont parmi les meilleures, mais aussi les plus contraignantes au monde. C'est pourquoi il est nécessaire, en parallèle, de renforcer le contrôle des importations. Il est également essentiel de lutter contre le recul du nombre de vétérinaires dans nos campagnes et de revaloriser les organismes gérant la sécurité alimentaire. Nous ne devons plus connaître de crises sanitaires, comme ce fut le cas Nous approuvons le maintien des mesures agroenvironnementales et climatiques. L'agriculture doit être écologiquement responsable et économiquement forte. Cette agriculture, notre agriculture, nous devons aussi la rendre attractive en mettant en lumière le savoir-faire de nos agriculteurs, en développant des circuits courts, qui répondent aux demandes des consommateurs, en soutenant la recherche et l'innovation, en valorisant des méthodes de production respectueuses de l'environnement, tout en assurant des rendements suffisants. L'installation des jeunes et la reprise des exploitations doivent aussi être un point essentiel. On constate dans certaines régions, dans la mienne par exemple, une réduction des surfaces agricoles. le fort développement des agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire conduit à une pression très forte sur les terres agricoles. La façade maritime et l'activité touristique associée contribuent également à la diminution de la surface agricole utile qui, forte de 457 000 hectares aujourd'hui, se réduit chaque année d'environ 2 500 à 3 000 hectares- il nous faut réagir. Nos agriculteurs participent activement à la revitalisation des territoires ; ils sont les premiers gestionnaires des ressources naturelles françaises. Concernant la politique forestière, nous regrettons qu'une trop grande dispersion des financements publics conduise à un manque de visibilité et

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous vivons aujourd'hui une période de transition de notre modèle agricole et de nos habitudes alimentaires. Nous ne devons pas rater ce rendez-vous et nous devons accompagner ces changements vers plus d'agriculture biologique et plus de sécurité sanitaire pour tous.

La balance commerciale continue aujourd'hui d'être excédentaire, et nous devons pérenniser cette situation par une montée en gamme de certains produits agricoles, pour obtenir, notamment, de meilleurs débouchés à l'international et assurer le développement d'une agriculture plus productive.

Il est devenu indispensable de produire une nourriture de qualité et dont le prix soit juste pour le producteur et l'acheteur. C'est

Ainsi, nous devons tenir compte du mal-être d'une trop grande partie de nos paysans et de nos pêcheurs, qui méritent comme les autres de vivre dignement de leur travail et de leur production. Au titre de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », le Gouvernement demande l'ouverture de 2,77 milliards d'euros en autorisations d'engagement de 2,86 milliards d'euros en crédits de paiement. Tout d'abord, la mission que nous examinons aujourd'hui doit se lire en parallèle avec la réforme fiscale prévue dans la première partie du projet de loi de finances pour Avec le Parlement, le Gouvernement souhaite, comme il s'y était engagé l'année dernière, simplifier les modalités de recours à l'épargne de précaution afin que les agriculteurs puissent faire face efficacement aux aléas de plus en plus importants auxquels ils sont exposés.

de budget que vous soumettez au vote du Parlement, monsieur le ministre, est cohérent et traduit une certaine stabilité par rapport au budget de l'année dernière, puisque celui-ci est sensiblement identique. Comme vous Comme vous avez déjà pu l'expliquer, la baisse de 500 millions d'euros correspond en grande partie aux allégements de charges sociales, qui sont passées sur le budget de la sécurité sociale, car il ne s'agit pas d'actions de développement agricole évidentes. Par ailleurs, la provision pour aléas sera ramenée de 300 millions d'euros à 200 millions d'euros, une baisse qui n'affectera pas le développement économique ni l'aide aux agriculteurs et à la transformation de l'agriculture, mais qui s'opère dans une période où nous sommes confrontés à plusieurs crises déclarées, notamment le phénomène de sécheresse, que je n'ai cessé de dénoncer ici même. En cas de nouvelles difficultés, vous vous êtes engagé, monsieur le ministre, à répondre de manière efficacement aux exploitants agricoles en difficulté.

Plusieurs mesures budgétaires, à l'instar de la loi ÉGALIM, viennent traduire le programme Ambition Bio 2022, présenté en juin dernier par le Gouvernement. Notons une augmentation pour la redevance pour pollution diffuse et le doublement progressif des moyens du fonds de structuration Avenir Bio, dont l'enveloppe sera portée de 4 millions d'euros aussi la subvention attribuée à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, l'Agence Bio, qui sera portée de 5,43 millions d'euros à 10,7 millions d'euros.

Par ailleurs, le budget alloué au secteur de la forêt et du bois bénéficie d'une augmentation substantielle de 250 millions d'euros. À ce budget de 4,6 milliards d'euros s'ajoutent évidemment les crédits de la PAC- plus de 9 milliards d'euros -et les allégements fiscaux. Cumulés, ce sont 23,4 milliards d'euros

traduit, conjointement avec la loi ÉGALIM, l'ambition d'une transition multiforme : une transition économique, avec l'inversion de la construction du prix, une transition écologique, en favorisant une agriculture moins consommatrice d'eau et de produits phytosanitaires. Comme le Président de la République s'y est engagé, la France sortira du glyphosate en 2021. Alors ça ...

Nous devons absolument combattre le développement d'une agriculture à deux vitesses : une agriculture sûre- bio, mais surtout peut-être plus onéreuse -et une agriculture pour les plus défavorisés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Ce désir de raboter en général tous les crédits des missions, comme vous le faites avec la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », ne passe plus auprès des agriculteurs. Dotée de 2,765 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 2,854 milliards d'euros en crédits de paiement, la mission que nous étudions aujourd'hui connaît une baisse de près de 17 %. Année après année, le constat amer est le même : vous tournez le dos à nos agriculteurs, aux consommateurs, à l'ensemble de nos concitoyens. Même si vous répétez inlassablement que la baisse du soutien à l'agriculture cette mission n'est qu'apparente, car elle est amputée des allégements de charges désormais intégrés au projet il n'en demeure pas moins vrai que cette baisse ne représente qu'un coût de 272 millions d'euros, et non de 552 millions d'euros comme c'est le cas actuellement Je l'ai dit, comme pour d'autres missions, le soutien de l'État passe de plus en plus par des allégements fiscaux et sociaux, aux dépens des soutiens aux crédits, qu'ils soient européens ou nationaux, et cela marque, de fait, le désengagement de l'État. Nous partageons d'ailleurs le constat des rapporteurs spéciaux, les dépenses de soutien aux exploitations agricoles, absolument nécessaires à la viabilité de nombre d'entre elles, demeurant sans tonus. Ainsi, tous les programmes connaissent des baisses, mais la plus forte est celle qui porte sur le programme 149, « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture », qui perd 154 millions d'euros. Pourtant, ce programme concerne les principaux dispositifs structurants de l'agriculture, notamment le cofinancement national des mesures de développement rural de la PAC : soutien à l'élevage dans les zones soumises à des contraintes naturelles, installation des jeunes agriculteurs, accompagnement des projets d'investissement des exploitations agricoles, mesures agroenvironnementales. En entrant dans le détail des crédits, c'est moins 90 millions d'euros de crédits pour l'action n° 27, Moyens de mise en oeuvre des politiques publiques et gestion des interventions. Or cette action regroupe les moyens dévolus aux opérateurs tels que l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO, l'Agence BIO, FranceAgriMer, l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, l'Agence de services et de paiement ; la liste n'est pas exhaustive. C'est moins 8,4 millions d'euros pour l'action n° 06, Mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation, et moins 18 millions d'euros pour l'action n° 01, Moyens de l'administration centrale. Monsieur le ministre, c'est encore moins 8 millions d'euros pour les DRAAF, les C'est toujours moins ! Dès lors, comment croire que ce budget permettrait tout à la fois de mener des actions de développement agricole et d'assurer la préservation de l'environnement, la transition vers l'agroécologie, le développement du bio et la meilleure protection sanitaire possible ? Comment croire qu'il sera possible de toujours faire mieux avec moins, alors que notre agriculture est aujourd'hui sinistrée ! Comme cela a été souligné lors de nombreux débats, vous affichez sur tous les terrains une préoccupation environnementale, mais les actes ne suivent pas Ils sont même en parfaite contradiction. La transition, c'est le changement, mais vous supprimez les moyens humains, et ce à tous les niveaux, alors qu'ils sont indispensables pour accompagner les agriculteurs vers l'agroécologie.

Alors qu'il faudrait renforcer le soutien à nos filières, ainsi que les moyens attribués aux administrations de contrôle, c'est l'option inverse que vous choisissez ! Comment allons-nous, demain, contrôler les dizaines de milliers de tonnes supplémentaires de viande bovine importées du Canada, du Mercosur ou de la Nouvelle-Zélande ? Comment être sûr que ces viandes auront été produites sans antibiotiques, sans hormones, sans alimentation animale issue de sols traités avec du glyphosate ? D'ailleurs, l'actualité récente nous donne raison, puisque a découvert que 150 tonnes d'aliments contaminés par un OGM non conforme aux réglementations européennes à destination du bétail français ont été distribuées à trois fabricants et douze éleveurs. D'après des associations de consommateurs, vingt pays sont aujourd'hui touchés par ces denrées contaminées. Il faut absolument condamner le manque de traçabilité en Europe : il a fallu plus d'un mois et demi avant que les autorités ne se saisissent du problème et que la société incriminée puisse donner aux États les éléments nécessaires pour retracer les lots infectés. De quoi compliquer ce travail de traçabilité

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » connaissent une baisse de 16,5 % par rapport à 2018, diminution qui s'explique par deux facteurs

importantes dans un contexte budgétaire malheureusement contraint, comme vous le savez. Il est crucial de conserver les moyens de répondre à la situation encore bien fragile de nombreux exploitants. Ce budget a quatre objectifs : le soutien à l'agriculture complété par des cofinancements européens ; le renforcement de la prévention et de la gestion des risques sanitaires la formation des jeunes, au travers des moyens consacrés à l'enseignement et à la recherche, en particulier l'enseignement agricole dans toute sa diversité ; enfin, la transformation de l'agriculture par l'innovation et sa modernisation, notamment soutenue par le déploiement du volet agricole du Grand Plan d'investissement. J'ajoute que certains dispositifs du PLF traduisent déjà l'esprit de la loi ÉGALIM, récemment promulguée ; je pense, notamment, au doublement des crédits du À ce titre, il est absolument nécessaire de ne pas décevoir les espérances nées lors des états généraux de l'alimentation, qui doivent pleinement mobiliser le Gouvernement pour faire de la loi ÉGALIM un succès. Ce n'est pas encore gagné, monsieur le ministre Cela ne repose bien évidemment pas que sur l'agriculture biologique, cela va de soi. En effet, ce texte avait pour ambition première d'améliorer le revenu des agriculteurs. Il est important de rappeler que cela repose sur trois facteurs

La reconquête du revenu des agriculteurs ne peut se faire, à mon sens, qu'en combinant ces trois éléments. Je voudrais maintenant évoquer quelques points de ce budget qui me paraissent importants. Après la suppression programmée du dispositif TO-DE, les débats parlementaires et votre mobilisation ont permis de le maintenir à 1,15 % du SMIC.

J'avais alors en parallèle proposé un amendement de repli à 1,20 % du SMIC. Ce point d'équilibre a été adopté en séance publique par l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier. Néanmoins, la question de la pérennité de ce dispositif reste en suspens.

Par ailleurs, je veux revenir sur la réforme de la fiscalité agricole et, plus particulièrement, sur les dispositions fiscales favorisant l'épargne de précaution, qui permettront à nos agriculteurs de mieux faire face aux situations et d'amortir les aléas, qu'ils soient climatiques, sanitaires ou de marché. Je ne puis que saluer la création d'un tel dispositif, longtemps attendu par la profession, à la fois simple dans sa mise en oeuvre et adapté à la situation de chacun. de budget met aussi l'accent sur l'installation et le soutien au renouvellement des générations, un soutien fondamental. Enfin, concernant la filière bois,

C'est pour cette raison que je soutiens pleinement l'amendement déposé par notre collègue Anne-Catherine Loisier, pour orienter la taxe carbone, afin de soutenir les investissements nécessaires dans la filière.

aux nouveaux défis de l'agriculture et de la forêt, mais également à la nécessaire transition énergétique, un domaine fort mal accompagné actuellement, je tiens à le dire, par le ministère de la transition écologique. Nous devons absolument privilégier une écologie de projets et non pas une écologie d'interdiction, perçue comme étant punitive. Monsieur le ministre, vous aspirez à ce que la France soit « souveraine d'un point de vue alimentaire » et que « son agriculture rayonne dans le monde

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens, tout d'abord, à féliciter les rapporteurs spéciaux et pour avis de l'excellence de leur travail. J'illustrerai leurs interrogations en évoquant deux points la situation de la filière fruits et légumes, ainsi que les conséquences du Brexit sur notre agriculture et la pêche. La filière fruits et légumes est l'une des plus fragiles de nos productions agricoles, car elle dépend fortement non seulement du contexte climatique et météorologique, mais également de la compétition internationale. Avec 388 000 hectares cultivés en fruits et légumes, 5,5 millions de tonnes, la France est le troisième producteur de l'Union européenne, loin derrière l'Italie et l'Espagne.

saisonniers bénéficient d'une réduction de cotisations patronales sur les contrats par le biais d'un dispositif spécifique que nous connaissons tous et que vous connaissez aussi, monsieur le ministre, les TO-DE. Nous avons été nombreux à vous alerter sur ce point, car nous craignons que, sous couvert d'économies budgétaires, les mesures que le Gouvernement propose ne viennent directement affecter la compétitivité de notre économie agricole. Le coût de la main-d'oeuvre française est déjà bien plus élevé que chez nos voisins allemands et italiens, à savoir respectivement de 27 % et 37 %. Il ne faudrait pas encore l'aggraver. En outre, ce secteur est directement affecté par les aléas climatiques, ceux qui sont liés à l'eau, c'est-à-dire les inondations et la sécheresse. Nous pensons qu'il est nécessaire de revoir la loi sur l'eau, pour faire évoluer nos capacités à créer et à gérer la ressource, tout en continuant à la protéger. Ces difficultés, particulièrement accrues pour la filière fruits et légumes, entraîneront une perte de souveraineté alimentaire pour notre pays. Or je sais votre attachement à celle-ci, monsieur le ministre, comme d'ailleurs à notre agriculture et à nos agriculteurs. à nos agriculteurs. En outre, j'évoquerai les conséquences du Brexit sur notre pays dans le domaine de la pêche maritime. Après un an de négociations, l'Union européenne et la Grande-Bretagne ont fini par s'entendre sur un projet d'accord de retrait. La politique européenne en matière agricole est essentielle pour la France. Les aides de la PAC représentent près des deux tiers des concours publics à notre agriculture. Nous devons être très vigilants à leur évolution dans la nouvelle politique PAC, mais aussi dans les conséquences du retrait britannique. Le Conseil européen a adopté dimanche dernier un texte réglant les relations avec Londres pendant une période de transition, qui pourrait se prolonger jusqu'en 2022. Cet accord, qui contient un volet sur les questions de pêche, prévoit un accès aux eaux territoriales britanniques, et les Britanniques resteront soumis aux quotas de pêche européens pendant la période de transition. Néanmoins, il faudra conclure un accord au plus tard d'ici à la mi-2020 pour régler cette question. Nous pouvons nous associer avec d'autres États membres comme les Pays-Bas pour faire valoir notre position. Je crois que la négociation pourrait se fonder sur les principes d'accès réciproques et sur le maintien des quotas existants.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Ferme France contribue à la richesse de notre pays, avec une balance excédentaire de 6 milliards d'euros, mais celle-ci s'érode d'année en année.

Personne ne l'ignore : nous ne vivons pas dans un bocal. Des pays émergents le sont de moins en moins et deviennent des puissances à part entière. L'agriculture française cherche à s'adapter à la mondialisation des échanges, et ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux de l'agriculture de demain. Bien qu'ils soient en permanence pointés du doigt comme de « présumés pollueurs », les agriculteurs se sont engagés dans la transition écologique en menant des actions concrètes. Ce qu'ils contestent, ce sont les calendriers et les moyens d'accompagnement mis en oeuvre, qui ne tiennent absolument pas compte de leur situation économique actuelle. Face aux phénomènes climatiques, la question de l'efficience des assurances récoltes et les modalités de l'épargne de précaution sont également des sujets importants pour aider les professionnels à surmonter ces épreuves, et ce dans des délais raisonnables. Depuis 2014, nous n'avons cessé d'intervenir sur la récurrence des retards d'instruction des aides du second pilier. La situation financière des exploitants ne peut supporter de nouveaux dysfonctionnements. Les propositions de la Commission européenne dans le cadre du Brexit et de la nouvelle PAC sont, vous le savez, inadmissibles. Sur la question des TO-DE, vous avez indiqué que l'Assemblée nationale aurait le dernier mot- cela tombe bien monsieur le ministre, le Gouvernement y dispose de la majorité ! Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir défendre nos exploitants. À titre d'exemple, je puis vous dire que les Bouches-du-Rhône doivent faire face à la concurrence italienne, espagnole, marocaine, où le coût du travail est nettement inférieur.

On évoque souvent le souvenir d'un arrière-grand-père exploitant. Parfois, on va jusqu'à parler d'une jeunesse passée à la campagne ... Permettez-moi de vous le rappeler, monsieur le ministre, en amour comme en politique, il n'y a que les actes qui comptent

Nous n'avions pas su alors trouver les nouveautés répondant aux grands enjeux que l'agriculture française doit relever et nous étions abstenus en considérant que l'essentiel restait à faire. Vous nous avez dit que le budget que nous examinons aujourd'hui, monsieur le ministre, n'était pas le vôtre, mais que vous le défendriez pleinement, ce qui est bien normal. Le revenu des agriculteurs, l'accompagnement de la transformation agroécologique des exploitations, la compétitivité des filières, la gestion des risques, l'approche de la future PAC : c'est à l'aune de ces enjeux que ce budget doit être apprécié. Au cours de l'année écoulée, à partir de l'initiative positive des États généraux de l'alimentation, les qualité de l'alimentation et des plans de filières. La loi a été promulguée, les ordonnances sur les seuils de revente à perte et les promotions sont prises, les négociations commerciales sont en cours. Pourtant, le doute persiste dans la profession même quant à l'efficacité de ces dispositifs. Tout en partageant les objectifs nous étions sceptiques au sortir de la discussion de cette loi. Nous le sommes toujours et d'autant plus que 1 million d'euros seulement sera consacré à son accompagnement.

La compétitivité des filières concernées ne s'en portera que mieux dans un contexte, vous le savez, où la concurrence sur les coûts fait rage. La transition agroécologique vers des produits de qualité à prix abordable en sera aussi facilitée. La sortie injuste et injustifiée à ce jour de certains territoires ancestraux de polyculture-élevage des zones défavorisées conduira aussi à des pertes de revenus importantes et à l'arrêt d'exploitations, voire pire. Ce sera le cas dans le Gers pour près de 110 éleveurs, dans l'Aude, dans les Deux-Sèvres, ainsi que dans d'autres départements. On ne peut l'admettre quand on connaît les territoires concernés, les hommes et les femmes qui y vivent avec autant de peine que de dignité

Monsieur le ministre, indépendamment de la diminution d'environ 300 millions d'euros de ses crédits, à périmètre constant, et malgré des mesures bienvenues en matière fiscale, ce budget 2019 ne prend pas, ou pas assez, en compte les grandes difficultés des filières,

qui ne nous convainc absolument pas sur le fond, certains de nos amendements, pourtant importants, car ils permettaient de prendre en compte les problèmes de nombreux agriculteurs, n'aient même pas pu être discutés. Et je reconnais volontiers, monsieur le ministre, que ce n'est pas de votre fait. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout le monde l'a dit : le budget alloué à l'agriculture n'est pas à la hauteur des enjeux et ne correspond aux besoins ni de l'agriculture ni des agriculteurs français. Pourtant l'agriculture va mal ! Je voudrais, au moment du vote de ce budget, que l'on n'oublie pas les premiers intéressés : un tiers d'entre eux ne gagne pas la moitié du SMIC,

vous le savez tout autant que moi, monsieur le ministre, ils subissent une administration omnipotente, qui n'est même plus capable de gérer les règles qu'elle a fixées

il va falloir apporter un certain nombre de réponses : des réponses pour mettre une barrière à la concurrence des produits qui ne respectent pas les normes françaises et élaborer une loi-cadre pour l'agriculture française, qui fixerait les règles du jeu entre les agriculteurs et les consommateurs français.

Vous ne devez pas les décevoir

devait être la « première étape d'une transformation sans précédent de l'agriculture française ». En jetant un oeil dans le rétroviseur sur les avancées engrangées depuis ce budget, on se dit que, à ce rythme-là, la transformation prendra du temps

atténuation du changement climatique, garantie d'une alimentation saine et suffisante, développement rural plus inclusif. Si vous souhaitez réellement aller vers une transformation sans précédent de notre agriculture, c'est sur la voie étroite, certes, mais praticable que ces organismes décrivent, qu'il faut vous engager. Or ce budget semble s'inscrire dans la stricte lignée du précédent : nous n'y trouvons ni les réponses aux grands enjeux de demain ni les solutions aux problèmes d'aujourd'hui. L'urgence, nous le savons tous, est de garantir un métier rémunérateur aux agriculteurs. Comme l'a justement souligné Franck Montaugé, la question du revenu est l'un des principaux motifs de déception de la loi ÉGALIM, après l'espoir qu'avaient suscité les États généraux l'année dernière.

Vous nous aviez répondu que, bien qu'il soit sympathique, le dispositif que nous adoptions ne pourrait pas tenir à l'Assemblée nationale. Et plutôt que d'essayer de convaincre les députés de ce que les sénateurs vous avaient fait remonter

cet anglicisme n'est évidemment pas de moi -, vous devriez peut-être commencer à le faire quand vous êtes face aux députés de votre majorité, qui semblent bien mal connaître l'agriculture française nous vous ferons objectivement des propositions concrètes et pragmatiques pour améliorer la situation économique de nos exploitations.

les restes à payer des prêts bonifiés supprimés en 2017 ! Aussi la diminution de 1,3 million d'euros en autorisations d'engagement marquerait un coup d'arrêt pour l'année prochaine. Cumulée à celle de l'année précédente, elle correspondrait à une baisse de 3,8 millions d'euros en deux ans, soit 7 % de moins par rapport à 2017. L'installation et le renouvellement des générations sont des problématiques majeures quand il est question de l'avenir de notre agriculture. C'est pourquoi il faut absolument maintenir les efforts financiers dans ce domaine. Il manque dans ce budget des mesures volontaristes pour répondre aux difficultés de trésorerie que connaissent de nombreuses exploitations. Aussi,

Ces derniers temps, les préoccupations de nos concitoyens en matière de qualité et de sécurité alimentaires, ainsi que leur attention à l'impact environnemental de ce qu'ils consomment, se font plus fortes que jamais.

très peu de positif et une grande déception. Le monde agricole a des défis à relever, chacun en convient. Or les actes ne sont pas à la hauteur des engagements pris. je voudrais manifester ma préoccupation et mon inquiétude pour la dotation de réserve pour aléas climatiques et problèmes sanitaires, qui est en baisse de 100 millions d'euros. L'enveloppe diminue malgré les difficultés actuelles. Les aléas sont de plus en plus fréquents et importants c'est le cas cette année avec la sécheresse, qui va causer de lourds préjudices. Il est regrettable que la ligne ouverte en 2018 ne serve pas à accompagner les éleveurs, qui subissent de plein fouet les effets de la crise. Une grande partie de l'agriculture française sinistrée par la sécheresse doit faire face à une situation sans précédent. Certes, comme vous l'avez dit en commission, monsieur le ministre, des aides exceptionnelles sont prévues, les compensations versées seront-elles à la hauteur et dans quel délai ? Pour certains départements comme le Jura, par exemple, la première coupe de fourrage a été correcte

Nos rapporteurs estiment d'ailleurs à juste titre que cette provision est un alibi, qui vise à masquer des coupes budgétaires. En 2018, quelque 94 % des dépenses de la réserve ont servi au paiement des refus d'apurement communautaire. Cette réserve de crise est en réalité une auto-assurance de l'État financée par des économies réalisées au détriment des agriculteurs. Voilà la vérité je souhaiterais que vous rassuriez nos agriculteurs, de plus en plus confrontés aux aléas de toute nature. Notre agriculture est soumise également à des risques sanitaires, comme, en ce moment, le risque de propagation de la peste porcine. Hélas, ce n'est pas la pose de clôtures électriques de part et d'autre de la frontière qui arrêtera le virus ! On voit ici que la notion d'aléa va devenir de plus en plus cruciale. En lien avec les problèmes sanitaires, je souhaiterais soulever le problème des déserts vétérinaires. En effet, les futurs vétérinaires choisissent de plus en plus fréquemment les soins pour animaux domestiques, délaissant la pratique en élevage. Que prévoyez-vous, monsieur le ministre, pour lutter contre ce phénomène ? Il faut conclure, ma chère collègue. Nos agriculteurs travaillent dur pour nous nourrir et assurer notre indépendance alimentaire. Ils méritent notre reconnaissance et notre soutien. Les crédits de la mission qui sont présentés aujourd'hui ne me paraissent pas à la hauteur des enjeux agricoles à venir. Aussi je ne voterai pas ces crédits, monsieur le ministre

parallèlement, les collectivités locales se sont mobilisées pour leur apporter des concours financiers. On voit bien que les dispositions prises vis-à-vis de l'agriculture par le ministère, que ce soit l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti fonds de garantie des calamités agricoles, ne sont que des palliatifs par rapport à une crise structurelle. Monsieur le ministre, le Président de la République a fait une déclaration importante,

Je ne laisserai jamais traiter un paysan d'empoisonneur ! Je me suis rendu à Rethel, dans les Ardennes, pour rouvrir un abattoir. Je n'ai pas peur de dire que nous avons besoin d'une filière d'élevage et d'abattoirs qui fonctionnent bien, en toute sécurité.

Elles favorisent aussi l'installation des jeunes agriculteurs, ce qui n'est pas négligeable. Désormais, ces aides sont intégrées, au niveau de leur financement, dans le Grand Plan d'investissement évoqué par le ministre. Toutefois, ce plan n'est pas encore réellement mis en oeuvre. Les moyens débloqués en 2019 apparaissant encore faibles, à savoir 158 millions d'euros en autorisations d'engagement et 216 millions d'euros en crédits de paiement, sur les 5 milliards d'euros annoncés sur la période 2018-2022. Il nous apparaît donc nécessaire, dans un premier temps et, de maintenir les autorisations d'engagement à un niveau similaire à celui de 2018. Je rappelle que, en 2017, les autorisations d'engagement pour le PCAE s'élevaient à 84,5 millions

c'est sans parler des prestations pour services environnementaux. Je ne les ai pas évoquées en discussion générale, mais elles le seront dans le cadre de la future PAC et pourraient permettre à l'agriculture française d'être reconnue pour tout ce qu'elle apporte à la société, dans son ensemble

Je vais vous en donner les raisons, moi qui ai fait de mon département, pendant une quinzaine d'années, le premier département « bio » de France, avec 50 % de produits bio proposés dans toute la restauration collective. Si le premier signe que l'on donne

confèrent les lois dont nous disposons. Avec Bernard Buis, mon collègue sénateur, que je salue bien volontiers, puisque c'est la première fois que je le rencontre dans cet hémicycle,

scolaire- l'enjeu est très important, puisqu'il s'agit de nos enfants -, nous devons absolument faire en sorte que les collectivités soient accompagnées de manière significative et très concrète. concrète. Ceux qui gèrent les restaurants collectifs peuvent être démunis, être freinés de multiples façons : il faut donc absolument débloquer ces situations. Les choses ne sont pas simples, nous le savons tous : il faut chercher des producteurs locaux,

une concurrence entre les ports européens pour recueillir une partie du flux des marchandises qui arriveront en Europe. Je sais aussi que les ports français n'ont pas été très bien traités jusque-là, en particulier les ports normands et

C'est ce que l'on fait quand on gère correctement une collectivité locale. Deuxièmement, nous ne sommes pas sûrs que le Brexit ne soit pas un Brexit dur le 31 mars 2019.

Pour mémoire, le gouvernement précédent avait porté les autorisations d'engagement concernant ces installations à 40 millions d'euros. M. le ministre évoquera peut-être le Grand Plan d'investissement avec ses 5 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros permettra des garanties la Banque européenne d'investissement pour l'installation des jeunes agriculteurs.

est non seulement vieillissante, notamment chez les agriculteurs, mais en baisse. Nous perdons 1 000 habitants par an pour une population de 170 000 habitants. Dans nombre de nos communes, les quelques agriculteurs restants sont trop souvent sans successeur.

Or l'Observatoire national démographique de la profession vétérinaire pour 2017 craint une diminution importante de ses effectifs. L'activité principale de ceux-ci s'oriente de plus en plus vers les filières « animaux de compagnie Ce phénomène pourrait s'aggraver dans les années à venir, à mesure que les jeunes praticiens ne remplacent plus les anciens vétérinaires ruraux, qui étaient proches de la retraite, pour se concentrer sur les soins d'animaux de compagnie dans les centres urbains. C'est un drame, mais tout comme ont surgi les « déserts médicaux », les premiers « déserts vétérinaires » sont apparus en France et devraient se multiplier d'ici cinq à dix ans dans certaines régions rurales. n'ignorez pas non plus que cela constituerait un drame pour nos territoires ruraux, pour notre élevage, ainsi que pour la sécurité sanitaire de la France dont nous parlons jusqu'à présent. Pour autant, certaines solutions ont fait leurs preuves. C'est le cas des « stages tutorés en milieu rural », financés par le programme 206, monsieur le ministre, Lors de leur dernière année du cursus des écoles nationales vétérinaires, les étudiants peuvent réaliser un stage tutoré. Une vingtaine d'entre eux a bénéficié de ce dispositif

Prenons l'exemple du Royaume-Uni, qui, pendant une certaine période, a dénaturé complètement les services sanitaires vétérinaires.

Les PAT sont des solutions intéressantes et pragmatiques pour consolider les filières sur un territoire dans le but de structurer la production, d'aider la structuration des marchés de gros, par exemple, et de mieux répondre à la hausse de la demande de la restauration collective.

cet amendement, nous tirons les conséquences de l'adoption au Sénat, le 1 février 2018, de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. Il s'agit de prendre en charge la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.

Monsieur le ministre Stéphane Travert, il me semble, avec tout le respect que j'ai pour vous, que vous apportez à une question politique et sociétale portée par nos concitoyens, une réponse administrative et technocratique. Considérant le débat que nous avons à l'instant, le Sénat semble s'orienter vers un vote très majoritaire. Aussi, parfois le Gouvernement doit écouter le Parlement. Monsieur le ministre, vous comprendrez que nous n'attendons donc rien d'autre que votre plein et entier soutien à notre amendement, qui vient répondre à une attente sociétale forte et vient traduire une prise de position claire et ferme de la Haute Assemblée, quels que soient les bancs politiques. Nous le répétons, il s'agit de protéger et de défendre les malades, au premier rang desquels les agriculteurs. Ces derniers sont en effet trop souvent montrés du doigt pour l'utilisation de ces produits, alors qu'ils sont, dans le même temps, les premiers et les plus nombreux à souffrir de leur effet nocif. Monsieur le ministre, je le répète, je compte sur votre constance pour apporter un soutien à notre amendement, conformément au vote que vous avez exprimé en février et juillet derniers au Sénat, et à la nécessité, comme vous le disiez si bien vous-même lors de l'examen de la loi ÉGALIM, que le Gouvernement écoute le Parlement.

Je mets aux voix l'amendement n° II-107 rectifié. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission des affaires étrangères et de la défense, ce budget constitue la première année de la mise en oeuvre de la loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025, qui a été adoptée il y a quelques mois. Le montant des crédits de paiement, hors pensions, inscrits dans le présent projet de loi de finances- 37,9 milliards

entre 2019 et 2023 soit inégalement réparti, avec une marge plus importante, qui ne pourra être gravie qu'en 2023, soit au début du prochain quinquennat et de la prochaine mandature. S'agissant des effectifs, les engagements sont également tenus, avec la création de 450 emplois. La répartition de ces postes est également conforme à la loi de programmation militaire, la majorité d'entre eux étant consacrée au renseignement et à la cyberdéfense. Toutefois, je m'inquiète de la sous-consommation des crédits du titre 2 en 2018. Cette dernière, qui est de 155 millions d'euros, illustre les difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels. Dans ce contexte, je me félicite du financement de mesures de revalorisation salariale et de la montée en puissance du plan Famille. Doté de 57 millions d'euros en 2019, contre 22,5 millions d'euros en 2018, ce plan comporte 46 actions relatives à la mobilité, au champ social ou encore à l'hébergement.

En 2019, les crédits de maintenance progressent de 7 % en autorisations d'engagement et de 12 % en crédits de paiement. Sur la durée de la programmation, 13,5 milliards d'euros devraient être consacrés aux infrastructures. Il s'agit là d'un effort important, important, qu'il me plaît de souligner, même si, selon les armées, il manque encore 1,5 milliard d'euros. L'entretien programmé des matériels progresse de 4,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement, pour accompagner la réforme du maintien en condition opérationnelle aéronautique.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, en contradiction totale avec l'article 4 de l'actuelle loi de programmation militaire comme avec l'article 4 de la future LPM, la solidarité interministérielle ne jouera pas. Ce renoncement aux principes augure mal de l'application de la future loi de programmation. Comment croire

Nos militaires ne choisissent pas de partir au front au péril de leur vie. La solidarité interministérielle témoigne, à leur endroit, de la reconnaissance de la Nation tout entière.

a le pouvoir d'engager nos forces, au nom de la France, sans passer devant le Parlement. Il est donc logique que sa décision trouve une traduction solennelle impliquant l'ensemble de l'action gouvernementale.

: « [ ...] Nous venons ensemble d'envoyer à nos armées un message clair : les privations sont finies, le renouveau commence.

Malgré les allégations du Premier ministre, cette décision aura, tôt ou tard, des conséquences sur le paiement de nos commandes et sur les livraisons elles-mêmes. Le deuxième message s'adresse au Gouvernement, et singulièrement à Bercy. Nous refusons de cautionner un budget qui compromet, dès son entrée en vigueur, la bonne exécution de la

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, M. Cédric Perrin, rapporteur pour avis, avec moi, du programme 146, « Équipement des forces », ne peut malheureusement être des nôtres aujourd'hui, en raison du décalage de l'examen de la mission « Défense ». Il m'a demandé de bien vouloir vous livrer son intervention. Madame la ministre, les crédits du programme 146 doivent augmenter sensiblement en 2019 : nous nous en réjouissons, en raison du caractère stratégique de ce programme, qui représente 30 % des crédits de votre ministère.

Elle permettra l'acquisition de nombreux matériels. Je salue notamment la poursuite du redressement des capacités de transport aérien, avec un A400 M Atlas, un MRTT Phénix deux C 130 J.

ou FREMM, 50 postes de tir du nouveau missile moyenne portée, ou MMP, et 89 blindés multirôles lourds Griffon. à m'arrêter un instant sur ce programme Griffon. En effet, à plusieurs reprises, lors de nos auditions en commission, nous avons demandé si le calendrier établi serait tenu. Nous avons reçu des réponses rassurantes, ce qui ne nous empêche pas de rester vigilants au sujet de ce programme emblématique.

en soit, l'entrée en LPM est fragilisée par les conditions de la fin de gestion de l'exercice 2018.

Il n'y a pas de miracles : ces millions d'euros, annulés aujourd'hui, devront être payés plus tard, c'est-à-dire au cours d'une LPM qui, avant même son premier jour, est plongée dans le rouge. Nous voyons malheureusement le redressement annoncé se heurter d'emblée à des logiques budgétaires qui, en définitive, posent la question des priorités politiques.

le problème n'est pas votre budget ou vos orientations, lesquelles sont conformes à la loi. Le problème vient de l'annulation, imposée par Bercy, de 404 millions d'euros dans le cadre du

la provision pour OPEX ne sera encore que de 850 millions d'euros. Bercy compte-t-il continuer l'an prochain à refuser d'appliquer la LPM que vous avez conçue et qui a été signée par le chef de l'État le 14 juillet dernier

C'est ce comportement court-termiste que nous espérions avoir dépassé avec la nouvelle LPM. Pour résumer, madame la ministre, qui prendra la décision relative à l'exécution du budget de la défense pour 2019 ?

? Madame la ministre, vous avez fait reposer une part importante de la LPM sur les coopérations européennes. À ce titre, nous vous avons fait part de nos préoccupations. Certaines informations récentes nous inquiètent tout particulièrement au sujet du partenariat franco-allemand. Saurez-vous nous rassurer sur ce point ? souhaiterions obtenir, sous forme de rapport, des informations détaillées quant à l'avancement des différents projets de coopération européenne en matière d'armement. Pouvez-vous également nous exposer ce qui, dans le budget pour 2019, traduit concrètement l'accélération des coopérations européennes que vous espérez ? Enfin, je tiens à évoquer un dernier sujet. Nous aimerions obtenir des éléments de comparaison à propos des coûts d'acquisition et d'entretien de nos matériels, par rapport à ceux que connaissent nos alliés européens et otaniens. La LPM prévoit que nous augmentions fortement les crédits d'équipement des forces. Il nous revient aussi de nous assurer que ces fonds supplémentaires profitent pleinement, et surtout principalement, à nos forces armées. La parole

Le programme 178 voit ses crédits de paiement augmenter de 8,9 % par rapport à 2018, pour s'établir à 8,78 milliards d'euros. Cette progression bénéficie au financement des opérations extérieures, lequel obtient 195 millions d'euros supplémentaires pour atteindre 600 millions d'euros. Si notre commission a soutenu la poursuite du « resoclage » budgétaire des surcoûts des OPEX, c'était à la condition que l'enveloppe globale des crédits de la mission soit augmentée à due proportion. Or tel n'est pas le cas. de loi de finances pour 2019 consacre aux OPEX sont encore largement insuffisants. Dans ce contexte, notre commission, qui a modifié l'article 4 de la LPM pour prévoir le financement interministériel des surcoûts dus et la proportionnalité de l'effort consenti par la défense, recommande vivement que cette disposition soit bien appliquée en 2019. L'allocation de 375 millions d'euros supplémentaires en faveur de l'entretien programmé du matériel, en 2019, est un effort nécessaire au regard des besoins immenses

de la disponibilité technique opérationnelle, la DTO, et maîtrise des coûts de maintenance. Il conviendra également de veiller au maintien des compétences en régie de l'État et des possibilités de mise en concurrence ultérieure. commissaires se sont abstenus de voter les crédits de la mission pour marquer leur mécontentement face aux décisions d'exécution pour 2018,

les jeunes équipages de l'armée de l'air peinent à se qualifier, alors que l'entraînement est un enjeu majeur de la marine. Enfin, Sentinelle pèse sur la capacité d'entraînement de l'armée de terre ; ne serait-il pas temps de définir Sentinelle 3 ?

avis. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, en tant que rapporteur pour avis du programme 212, je prends acte de l'augmentation modérée des crédits de titre 2, laquelle est de

sont désormais bien connues -, sans oublier un renfort opérationnel au profit de la marine et de l'armée de l'air. Cette hausse des crédits de titre 2 permet, en outre, de financer un plan catégoriel d'envergure, d'envergure, qui autorise enfin la mise en oeuvre de la seconde annuité du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », suspendue l'année dernière par mesure d'économie. Cette décision nous avait préoccupés. En effet, nous sommes attachés à ce que la transposition en faveur des militaires des mesures affectant la rémunération des fonctionnaires civils soit assurée sans retard, afin d'éviter que des écarts, ressentis comme inéquitables, ne se creusent au détriment le plan catégoriel comporte diverses mesures de revalorisation salariale et indemnitaire, notamment en faveur des praticiens des armées et, plus largement, au bénéfice des métiers sous tension, notamment la création d'une nouvelle prime de lien au service. à se substituer à cinq primes existantes. Elle est conçue comme un outil plus souple, à la disposition des différentes armées. Elle a vocation à favoriser l'attractivité des emplois de la défense, la fidélisation de ses personnels et la valorisation de ses compétences critiques. Il s'agit là- on le sait -d'un enjeu crucial pour les armées. Leur modèle de ressources humaines « à flux » impose un constant renouvellement des effectifs. Dans le même temps, elles doivent attirer des compétences rares et recherchées dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Pouvez-vous nous éclairer au sujet de la méthode et du calendrier ? De plus, la perspective de la réforme des retraites suscite des inquiétudes dans le monde militaire. La réforme s'accommodera-t-elle du maintien de ces dispositions, qui mettent en jeu la pérennité du modèle de ressources On pense, bien sûr, aux bonifications de cotisations liées à l'activité opérationnelle, à l'existence d'une pension à liquidation immédiate, ou encore aux limites d'âge basses, qui sont liées aux carrières courtes des militaires. En d'autres termes, pouvez-vous nous certifier que la singularité militaire sera bien prise en compte à l'occasion de cette réforme ?

effet, 1,5 milliard d'euros d'investissements ont été reportés au-delà de 2025 ; d'autre part, la soutenabilité de la politique immobilière est incertaine, en raison de la saturation des services de soutien.

ce n'est pas difficile ... -en cas d'application de la décote : à défaut de recettes, le ministère doit bénéficier de logements. Je conclus en évoquant la cession du bâtiment de l'ancien hôpital du Val-de-Grâce.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le cadre budgétaire du programme 144 est, disons-le d'emblée, positif, car il respecte la trajectoire définie par la LPM, à savoir l'augmentation progressive des crédits d'ici à 2025. Les crédits d'études amont représentent, à eux seuls, un peu plus de la moitié des crédits du programme, et progresseront de 35 millions d'euros pour s'établir à 758,5 millions d'euros.

comme nos collègues rapporteurs pour avis du programme 146, nous sommes inquiets des conditions de la fin de gestion de 2018 : pour le programme 144, ce sont 20 millions d'euros qui sont annulés. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser où ces coupes seront concerne le soutien à l'innovation, qui constitue l'un des deux axes de ce programme, l'autre étant le renseignement, nous portons, globalement, une appréciation positive, du fait, non seulement, de la hausse des crédits, mais aussi de l'orientation que vous avez retenue, en soulignant à maintes reprises l'importance que vous accordez à l'innovation. Naturellement, il ne faut pas que ces mesures restent un effet de mode. Dans ce contexte, si nous ne voulons pas que notre industrie de défense, aujourd'hui, et nos armées, demain, connaissent le déclassement technologique, il faut redoubler d'efforts sur le front de l'innovation. Le

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la LPM a exposé clairement les menaces et les priorités. Dans un monde plus incertain et plus dangereux, la France doit poursuivre ses efforts dans le domaine du renseignement.

Ces difficultés de recrutement et de fidélisation, globalement, mais pas complètement surmontées par la DGSE, tiennent également aux singularités des profils recherchés, ainsi qu'à la faiblesse des viviers, notamment dans le domaine du numérique. d'un problème structurel, qui touche tous les secteurs de l'État. Il est regrettable que les écoles d'ingénieurs et les universités soient dans l'incapacité de répondre à la croissance des demandes, ce qui crée des tensions sur le marché du travail. Sans une politique active d'orientation vers les filières scientifiques, la France aura, à terme, des difficultés à suivre les pays concurrents ou adversaires dans le domaine du renseignement technique et de la cyberdéfense. C'est un véritable enjeu de sécurité nationale

de l'hétérogénéité et de la vétusté de nombre de bâtiments. Ils ne correspondent plus aux besoins et à l'activité de ces services et nuisent, en outre, à leur attractivité comme à la fidélisation de leurs agents. Les programmes de rénovation et de construction sont des opérations complexes la saturation des emprises oblige à rénover sans interrompre l'activité et les exigences de sécurité sont maximales. S'agissant de la DGSE,

La DRSD verra, en 2019, le démarrage du projet de restructuration du site central pour un coût évalué à 60 millions d'euros. un plan pluriannuel de rénovation des directions zonales et des postes sera financé pour un montant de 16,5 millions d'euros. Nous veillerons

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur

cela a été rappelé, 326 sénateurs ont voté ce texte. Nous avons adhéré à votre démarche d'une LPM « à hauteur d'hommes », qui se préoccupe des militaires et de leurs familles, et pas seulement des équipements. Nous avons soutenu les deux volets de ce texte, la réparation et la préparation de l'avenir, tous les deux indispensables. C'est pourquoi vous ne serez pas étonnée que je reconnaisse ici, tout d'abord, qu'il y a du positif dans le projet de budget pour 2019,

Les presque 700 millions d'euros supplémentaires sur les équipements doivent ainsi permettre de véritablement commencer le grand chantier de modernisation de nos armées. C'est votre combat, madame la ministre ; c'est aussi le nôtre Naturellement, il y a des points qui appellent une plus grande vigilance, notamment concernant les ressources humaines : la façon dont seront traitées les retraites des militaires, la mise en oeuvre de la nouvelle politique de rémunération,

en nouveaux fusils HK416, qui arrivent pourtant au compte-gouttes dans les régiments ! Au-delà de ces exemples éloquents, il y a plus grave : c'est le doute que ce mouvement soudain de pure logique comptable peut faire naître sur la détermination du Gouvernement à suivre la feuille de route, difficile, que trace la LPM. S'il faut déjà raboter près d'un demi-milliard d'euros, alors que la LPM n'est même pas encore commencée, comment ferons-nous lorsqu'il faudra ajouter chaque année un volume encore plus important de crédits au budget de la défense ? Le message adressé par le collectif budgétaire est désastreux, et tout cela laisse une immense impression de gâchis, quelques mois seulement après l'adoption presque unanime de la LPM. La confiance finira par laisser place au doute Madame la ministre, nous avons travaillé en responsabilité, vous et nous, sur la LPM. Nous ne remettons pas en cause votre bonne foi. Nous savons quel est votre combat, il est aussi le nôtre :

Sans cette initiative malheureuse sur le collectif budgétaire, nous aurions voté sans réserve le budget de ce premier exercice de la LPM, mais à cause de cela, une large majorité des sénateurs va s'abstenir. Nous manquons une belle occasion de rassembler à nouveau le Sénat derrière nos armées et aussi derrière vous, madame la ministre. Tout cela est bien dommage ...

et faire le contraire de ce qui est spécifiquement prévu dans la LPM ? J'ai lu avec attention la lettre que le Premier ministre a bien voulu m'adresser à la suite du communiqué de presse de notre commission.

C'est oublier que les moyens que nous avons décidé de consacrer à notre défense dans la LPM sont loin d'être un luxe ! Les défis sont colossaux, vous les connaissez comme moi, combler les lacunes capacitaires, moderniser les équipements, développer nos capacités de renseignement, remettre en état des infrastructures délabrées, investir les nouveaux champs de conflictualité, redonner de l'air au service de santé et au commissariat des armées et renforcer l'attractivité du métier des armes, à l'heure où la concurrence des recruteurs du privé menace les ressources humaines des armées. Oui, il y a aura besoin de l'effort prévu en LPM, et si Bercy persiste à venir chercher un demi-milliard d'euros, un milliard d'euros ou plus sur le budget des armées chaque année, cela ne fonctionnera entendu un argument assez troublant : quand le Gouvernement- pas vous, madame la ministre -affirme que les annulations de crédit n'auront aucun impact, que faut-il en conclure

Ne faut-il pas plus de subsidiarité pour les bases de défense ? Les commandants de base, eux, sauront engager les crédits au plus près des besoins, au lieu d'être corsetés pour commander un transport, gérer l'habillement ou la cantine ou repeindre un couloir ! Cette question d'organisation doit être traitée, au risque d'empêcher la remontée en puissance. La question des ressources humaines et des recrutements nous inquiète aussi : quelque 155 millions d'euros n'ont pas été dépensés sur le titre 2 cette année. Chacun connaît la difficulté de maintenir les compétences dans nos armées, vu le niveau des rémunérations et la comparaison avec ce qui a cours dans le Aussi, l'idée qu'il reste en fin d'année 155 millions d'euros non dépensés nous laisse songeurs. La centralisation de la politique des ressources humaines au niveau du secrétariat général des armées a-t-elle vraiment amélioré le pilotage de la masse salariale ? Ou, tout simplement, est-ce un mal plus profond, celui de la perte globale d'attractivité du métier des armes par la conjonction du surengagement et de la faiblesse des rémunérations ? Je ne doute pas, madame la ministre, que ce sont des questions sur lesquelles vous allez vous pencher de très près. Nous vous accompagnerons dans ces investigations. Ce que souhaite notre commission, vous le savez, c'est non pas l'échec du Gouvernement, mais la réussite de notre modèle d'armée, parce que cette réussite est la condition de la défense de la France et des Français.

Ce sont des projets concrets, qui contribuent à l'attractivité de la carrière militaire pour les jeunes, qui vont ainsi servir leur pays dans des conditions améliorées par rapport à ce qu'ont connu leurs aînés.

Nous savons tous par expérience à quel point ce service est une composante essentielle de la solidité et de la confiance de nos forces armées, et à quel point il constitue un pôle d'excellence dans la médecine française et la recherche.

madame la ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Défense » sont essentiels pour la préservation de notre sécurité et de nos valeurs, mais aussi de nos intérêts, du fait de notre présence sur l'ensemble du globe. Ces crédits doivent en priorité assurer la sécurité des militaires déployés dans le monde. Au moment où nous parlons, ils sont près de 5 000 au Sahel, où ils remportent chaque jour des victoires contre le terrorisme, plus de 1 000 au Levant, que ce soit en mer, sur terre ou dans les airs, pour lutter contre ce qui reste de Daech et 10 000 à assurer la présence et la souveraineté de la France de la France dans le monde. Ces crédits sont essentiels, enfin, car ils doivent contribuer à préparer l'avenir, en nous permettant d'investir dans l'innovation pour préserver notre liberté d'action et d'assurer notre capacité à dissuader tout adversaire potentiel. Jeudi dernier, le chef d'état-major de l'armée de l'air a notamment souligné son inquiétude face à la prolifération des systèmes d'anti-accès, qui mettent en péril notre supériorité aéronavale. Face à ces défis, nous avons deux préoccupations ; nous les avons déjà exprimées lors des discussions sur la loi de programmation militaire. Première préoccupation, le budget des armées doit être sincère. Certes, madame la ministre, j'entends l'argument d'une hausse sans précédent du budget de la défense depuis de nombreuses années,

Nous appelons à ce que le reliquat soit effectivement et concrètement assuré par la solidarité interministérielle, comme l'a indiqué Dominique de Legge, et non par le budget des armées.

L'année 2019 verra la création de 450 postes, en particulier dans les secteurs du renseignement et de la cyberdéfense. Nous comprenons ces priorités, mais nous souhaitons que les missions conventionnelles des armées reçoivent également le renfort humain dont elles ont besoin. À ce niveau, nous sommes confrontés à un fait préoccupant : une sous-consommation des crédits de personnel pourrait être constatée en 2018. Sommes-nous face à un creux conjoncturel ou à un déficit chronique d'attractivité de la part des armées ? Pourriez-vous, madame la ministre, nous éclairer sur ce point ?

Il faut placer les efforts de la Nation, comme vous le dites avec justesse, madame la ministre, « à hauteur d'hommes ». Sur le plan humain, nous avons d'autres questionnements. Le projet de service national universel, SNU, nous interpelle.

Le SNU devrait être expérimenté à l'été 2019. Or aucun crédit n'a été inscrit à ce titre dans le présent projet de loi de finances, ni sur le budget du ministère des armées, ni sur celui du ministère de l'éducation nationale. Nous craignons une déstabilisation de la LPM et nous demandons à être rassurés sur ce point. Pour permettre d'exercer pleinement leur métier, les hommes ont besoin d'équipements bien entretenus et renouvelés. En 2019, les crédits pour l'entretien programmé du matériel connaîtront une hausse exceptionnelle en autorisations d'engagement de plus de 4,6 milliards d'euros, ce qui représente un doublement. Cette augmentation concernera en particulier le maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et contribuera à la mise en place de la nouvelle direction de la maintenance aéronautique. Alors que se déroulait, la semaine dernière, le Forum Innovation Défense, il est évident que la capacité du ministère à investir dans les technologies de demain est indispensable à notre effort de défense. Nous saluons ainsi la hausse des crédits dédiés à la recherche et au développement, qui sera de l'ordre de 180 millions d'euros Toutefois, en matière d'effort d'armement et d'équipement, nous souhaitons rappeler notre vigilance quant aux mouvements de crédits en cours, qui peuvent parfois déstabiliser des programmes entiers. L'exemple du récent projet de loi de finances rectificative nous a montré à quel point ces budgets sont fragiles et soumis aux aléas budgétaires.

Le Parlement a voté une trajectoire budgétaire ambitieuse, la plus ambitieuse depuis de nombreuses années. Nous n'accepterons pas de la voir remise en question en permanence par des arbitrages de Bercy. Cette tension entre les ministères des armées et du budget doit cesser, si nous voulons assumer collectivement l'effort de défense que nous avons tous voulu. Je rappelle à ce titre que les plus hautes « marches » budgétaires ne doivent être gravies qu'à partir de 2023. Le plus dur est donc devant nous ! Un proverbe tibétain dit : « Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le vote des crédits de la défense est toujours un moment singulier, incontournable, car c'est un moment de vérité budgétaire et politique. C'est l'occasion de vérifier si le Gouvernement respecte ses engagements en allouant les moyens nécessaires à l'application de lois que nous votons. La question est simple : le budget des armées pour 2019 est-il en adéquation financière avec la loi de programmation militaire votée il y a quatre mois, après un vrai travail de concertation ? Madame la ministre, nous savons votre engagement personnel dans la recherche de crédits à la hauteur des ambitions françaises en matière de défense, ambitions imposées par nos responsabilités internationales et par une sécurité mondiale rythmée par une instabilité géopolitique croissante. Pour autant, madame la ministre, je suis au regret de vous dire que, malheureusement, votre détermination n'a pas suffi Ce budget devait incarner « l'antichambre » de la première année de la loi de programmation militaire. Or, une fois de plus, nous avons assisté au scénario « gel de crédits, dégel et crispation sur toutes les

Pourtant, vous nous aviez promis que l'heure était à la réparation et à la préparation de l'avenir. Ces annulations augurent mal de l'entrée dans la nouvelle LPM, alors même que la France n'a pas réduit la voilure des OPEX. De fait, la problématique du maintien en condition opérationnelle, ou MCO, reste centrale, car l'usure des matériels et la rudesse des théâtres exigent un rythme de remplacement plus soutenu. Il y va de la sécurité de nos soldats.

Que dire également de la fin de la solidarité interministérielle dans le financement des OPEX ? Que penser des déclarations du Premier ministre, selon lesquelles les armées peuvent assumer intégralement les OPEX ? Cela m'amène à deux remarques. La fin de l'interministériel, c'est la négation de la LPM. Est-ce là toute la considération pour le pouvoir législatif et la représentation nationale ? Ensuite, l'interministériel n'est pas uniquement une question comptable : c'est aussi un partage du coût de la sécurité et de la défense de la Nation entre tous les ministères. En termes symboliques, ce n'est pas un détail. Peut-être me répondrez-vous que des reliquats de crédits de personnel, à hauteur de 150 millions d'euros, permettront d'amortir ces annulations ? Malheureusement non, car cette non-consommation incarne parfaitement le défi de la politique de ressources humaines, auquel le ministère doit faire face : recruter, rémunérer et fidéliser. C'est particulièrement vrai dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense. Les, leur exploitation et leur protection représentent un enjeu économique primordial. En outre, comment être attractif dans un secteur où les salaires dépassent ceux des généraux ? Certes, la réserve citoyenne pourrait offrir un début de réponse, mais encore faudrait-il mieux recenser et utiliser les talents des réservistes. Madame la ministre, je profite de cet instant pour vous demander de nous éclairer sur l'état de la réserve citoyenne, qui pourrait être mieux utilisée, en particulier à l'étranger pour l'organisation de la Journée défense et citoyenneté. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour continuer sur les questions technologiques, je voudrais attirer votre attention sur l'importance de notre souveraineté

À l'heure où les « rançongiciels » se développent, nous devons réfléchir à l'utilisation des logiciels libres dans les services et par les opérateurs sensibles. La dépendance de la défense envers Microsoft, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'écrire, est un handicap, voire une menace pour cette souveraineté numérique que nous devons construire. À cet instant de la discussion et en dépit du constat négatif sur la réalité de votre budget et ses lourdes conséquences sur les armées, je voudrais, madame la ministre, vous remercier pour votre action vis-à-vis des soldats et de leurs familles. Il me paraît important de rappeler qu'il n'est point de défense sans ressources humaines. Certes, nous rendons très régulièrement un hommage appuyé et solennel aux hommes et aux femmes de la défense. Mais ces hommages et cette reconnaissance doivent se traduire par des actes. Nous ne pouvons donc que vous soutenir concernant le plan Famille mis en place l'année dernière et qui devrait monter en puissance. Il y a en effet derrière chaque soldat une famille pour qui le quotidien est souvent difficile. Madame la ministre, vous l'aurez compris, je suivrai, avec mon groupe, l'avis de la commission des finances, qui a conclu à une position de sagesse, sagesse responsable, mais empreinte de lassitude et de lourdes inquiétudes concernant l'environnement et toute la communauté de défense.

Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, il y a six mois, nous discutions de la programmation militaire 2019-2025. Lors de ce débat, notre groupe avait pointé une vive inquiétude quant au choix de reporter la majorité de l'effort de défense à la fin du quinquennat, voire après les élections de 2022. Autant dire notre attention sur ce premier budget post-LPM. Avant toute chose, il faut rappeler notre profond doute à l'égard de l'objectif des fameux 2 % du PIB de l'effort budgétaire de défense. Cet objectif appelle, selon nous, un débat démocratique qui n'a toujours pas eu lieu.

que nous avons un désaccord sur le financement des OPEX. La défense nationale concerne, selon nous, l'ensemble des acteurs publics de l'État.

selon moi, d'autant plus incohérent que le ministère de la défense participe lui aussi à ce fonds. Dans ces conditions, pourquoi ne pas prévoir une ligne budgétaire suffisante au sein du programme 178 ?

Je poursuis sur la question de l'immobilier. Les gouvernements successifs ont fait le choix de vendre le patrimoine de la défense, alors que les besoins étaient criants, du fait de la mobilisation toujours plus importante des effectifs et de la vétusté des locaux existants. Le plan Famille doit permettre de répondre, en partie, à cette problématique. Nous soulignons l'engagement dans ce budget de presque 2 milliards d'euros pour planifier les nombreuses améliorations et rénovations de bâtiments de défense. C'est une très bonne chose, madame la ministre Pour poursuivre, vous connaissez, mes chers collègues, notre désaccord sur l'augmentation des crédits apportés à l'OTAN, à hauteur de 84 millions d'euros sur le budget de la défense et de 28 millions d'euros sur le budget de l'action extérieure de l'État.

Comment construire une nouvelle politique de sécurité collective en Europe et non une Europe de la défense arrimée à l'OTAN ? Voilà la question dont nous devrions débattre. Autre point de désaccord, que j'ai également souvent évoqué ici, le plan de modernisation nucléaire, qui mobilisera 4,5 milliards d'euros. En consacrant toujours plus d'argent

J'insiste également sur la baisse des crédits de l'action sociale en direction des militaires. Il s'agit ici d'un message que nous aurions aimé différent. Les séquelles de sont encore très présentes- vous en êtes consciente, madame la ministre, je le sais.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, monsieur Christian Cambon, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis nos derniers débats, ici même, lors de l'examen de la loi de programmation militaire, la situation du monde ne s'est pas apaisée. La montée des menaces a été largement décrite dans la dernière Revue stratégique. La menace terroriste, si elle a été largement circonscrite par nos interventions, notamment avec les opérations Barkhane et Chammal, est toujours présente et engage nos forces armées en opérations extérieures et intérieures. Je tiens ici à saluer la détermination, le courage et le professionnalisme de tous nos soldats et de leurs chefs, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de la Marine. Au-delà des opérations extérieures, les Français les côtoient au quotidien et il n'est pas rare qu'ils les remercient ou les saluent avec admiration et bienveillance. Ils patrouillent chaque jour dans nos rues en s'intégrant parfaitement aux dispositifs mis en place de manière conjointe et coordonnée par l'ensemble de nos forces de sécurité. Certains d'entre eux seront sur tous les théâtres d'opérations lors des prochaines fêtes de fin d'année et, pour avoir partagé quelques réveillons à leurs côtés, je sais ce que cela représente pour leurs familles. Derrière chaque soldat, il y a des parents, des conjoints, des enfants. Il y a aussi, et je tiens à insister sur ce point, notre pays et ses valeurs, que nos forces armées servent sans hésitation, fût-ce au prix du sacrifice suprême. Je pense aussi à nos soldats blessés et aux familles endeuillées. Notre travail dans cet hémicycle doit prendre tout cela en considération au moment où nous débattons du budget de la défense. En ce sens, au Sénat, nous n'avons pas attendu les artifices de communication d'un soi-disant « nouveau monde » pour considérer que certains sujets revêtent une importance qui dépasse les oppositions classiques entre partis politiques et appelle une approche collective au-delà de toutes les travées, sans oublier nos différences et nos divergences qui enrichissent nos travaux. Notre défense appelle sérénité et efficacité. Vous avez pu, madame la ministre, constater l'an dernier, lors du précédent débat budgétaire et au cours de la discussion de la loi de programmation militaire, que le Sénat est un lieu de débat constructif et créatif. Le président Cambon a repris le flambeau de ses prédécesseurs et je tiens à le remercier, lui et l'ensemble de nos collègues, pour la qualité de nos échanges et de nos débats en commission. Ici, nous travaillons en confiance et avec vigilance. Nous jugeons sur pièces ! Lors de la loi de programmation militaire, vous avez proposé un cadre de confiance en positionnant les futurs engagements budgétaires à « hauteur d'homme » et en suscitant beaucoup d'espoir d'amélioration pour nos armées. Nous avons voulu croire aux promesses d'un effort inédit et d'une remontée en puissance exceptionnelle. Cette démarche s'inscrivant en continuité du travail impulsé par le précédent président de la République, François Hollande, notre groupe l'a soutenue tout en émettant des réserves quant à son exécution et à la traduction des paroles en actes. Or, dans les actes, la fin de gestion de l'exercice 2018 est marquée par la contradiction de l'article 4 de la loi de programmation militaire sur la solidarité interministérielle quant aux surcoûts des OPEX. Cette disposition primait jusqu'alors et jusque dans le texte que nous avons voté en toute bonne foi le 4 juillet dernier. Les 404 millions d'euros supportés en 2018 par le seul budget des armées seront répercutés dès 2019 et entament donc largement les promesses faites par l'actuel gouvernement à nos armées. La loi de programmation militaire n'est pas encore en oeuvre que ces engagements sont déjà remis en question. Ce n'est pas, comme nous l'avons entendu, une simple question de technique budgétaire. C'est un problème politique dont nous nous demandons quelles seront les répercussions concrètes. Ce problème politique vient ternir l'impression générale de l'augmentation de 4,2 % du budget de la défense pour 1,7 milliard d'euros, qui l'inscrit dans la trajectoire fixée par la loi rectificative pour 2018, le doute est là. Il ne permet pas d'être assuré, par exemple, que l'augmentation du programme 146 aura la portée escomptée et que l'ensemble des commandes et livraisons d'équipements seront au rendez-vous. La logique budgétaire qui s'est appliquée ces dernières semaines pour le budget de la défense, consistant à prendre plus au ministère des armées parce qu'il a été doté de plus de crédits, risque d'être démultipliée lorsqu'il s'agira de garder le cap et de gravir la dernière grande marche avec l'augmentation de 3 milliards d'euros annuels dans la seconde partie de la loi de programmation militaire. L'exercice de travaux pratiques et concrets risque de se heurter encore plus durement à la logique de Bercy. Cependant, dans ce contexte d'incertitudes, il y a tout de même des signaux positifs à saluer. L'aspiration profonde au sein de nos armées portant sur les conditions de vie apparaît néanmoins prise en compte. Je pense à l'augmentation des crédits pour le plan Famille, portés à 57 millions d'euros. Cela va dans le bon sens et nous soutiendrons toutes les décisions qui permettront de poursuivre cette dynamique. L'un des grands enjeux de ces prochaines années porte en effet sur les capacités de fidélisation des personnels de nos armées. Nous devons faciliter la vie de nos soldats, qu'ils soient sur base, en caserne ou en situation de mobilité. Trop souvent, les tracas du quotidien quant à la recherche d'une place en crèche ou d'un appartement viennent s'ajouter aux difficultés d'un métier soumis à une pression constante. Comme le relève le 11 rapport du Haut comité d'évaluation de la condition militaire de septembre 2017, le premier facteur de départ de l'institution militaire porte sur la conciliation entre vie privée et vie militaire pour plus de 55 % des militaires interrogés. Nous avons le devoir de mettre nos soldats dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en opération mais aussi en dehors. De ce point de vue, pourriez-vous, madame la ministre, nous éclairer sur les prochaines étapes du plan Famille et d'autres projets que le ministère serait amené à porter pour situer son action sur l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires À cet enjeu de fidélisation s'ajoutent d'autres enjeux en termes de ressources humaines, avec le recrutement de 6 000 personnels sur la période 2019-2025.

Ensuite, je repose la question des moyens et des dispositifs de recrutement et d'intégration dans un contexte où 62 % des militaires envisagent de quitter la fonction. Le plan Famille est un levier d'attractivité qui porte essentiellement sur les personnels déjà sous contrat, mais qui ne sera peut-être pas suffisant pour celles et ceux que nos armées souhaiteraient attirer. Dans la pratique, pour l'année 2019, ce projet de loi de finances 199 dans le renseignement et 107 dans la cyberdéfense, soit 68 % des postes créés. Si je tiens à saluer ces créations de postes, j'observe qu'il s'agit d'emplois faisant appel à un haut niveau de compétences et à des profils particuliers. Sur ces profils, le ministère des armées est en concurrence avec le secteur privé, qui bénéficie d'une attractivité plus importante et qui est, en tout état de cause, rompu à l'exercice depuis de nombreuses années. En conséquence, l'institution va devoir mettre en oeuvre une stratégie d'attraction des meilleurs profils. Je vous pose donc la question, madame la ministre : quelles mesures le ministère entend-il prendre afin d'attirer et d'incorporer ces hauts potentiels ?

Nous ne pouvons regarder ce budget « Défense » dans le projet de loi de finances pour 2019 qu'à travers un prisme de doutes et d'incertitudes, conséquences directes des conditions de fin de gestion de l'exercice budgétaire qui s'achève. Budget 2018 pour lequel vous nous annonciez « un budget sincère, contrairement », je vous cite, « aux gouvernements précédents ». L'impact de 319 millions d'euros annulés sur le programme 146 n'est pas encore mesurable concrètement en termes d'équipements, mais nous savons, par expérience, qu'il y aura des effets à moyen ou long terme. Ce n'est pas un bon signal dans la perspective du comblement de nos lacunes capacitaires. Ce n'est pas non plus un bon signal donné par le Gouvernement à l'aube de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de programmation militaire. Nous savons que nous n'avons pas besoin de vous convaincre, vous, madame la ministre. Cohérents avec ce que nous disons depuis votre entrée en fonctions consistant à soutenir les avancées au service de notre défense et à nous opposer aux reculs, nous allons envoyer, à notre tour, un signal au Gouvernement. En conséquence, le groupe socialiste et républicain s'abstiendra sur le vote des crédits de la mission « Défense ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les présidents de commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'affichage des mesures inscrites dans le budget 2019 vient valider les axes de réforme portés par la loi de programmation militaire dont notre groupe partage pleinement les ambitions. Il s'agit en effet du premier budget de cette loi de programmation militaire 2019-2025, que le groupe Union Centriste que je représente avait largement soutenue lors de son examen par notre assemblée. Avec une augmentation de 1,7 milliard d'euros de crédits par rapport à 2018, l'effort financier permet au budget d'atteindre 35,9 milliards d'euros, hors pensions. Nous sommes donc sur la bonne trajectoire pour atteindre notre objectif d'allocation de 2 % de la richesse nationale à notre impératif de défense. Je tiens tout d'abord à saluer, pour la première année, une remontée en puissance des effectifs au sein du ministère, avec la création nette de 450 emplois affectés principalement dans les domaines du numérique, du renseignement et de la cyberdéfense. Ce budget intègre ainsi deux axes structurants de la loi de programmation militaire, la préparation aux conflits du futur et l'innovation, avec, notamment, 758 millions d'euros prévus pour les études amont, soit une hausse de 5 % des crédits. À l'heure de révolutions numérique et sociétale, ces effectifs et ces crédits supplémentaires sont indispensables pour demeurer compétitifs et protégés face aux nouvelles menaces qui apparaissent autour de nous. Les nouvelles technologies constituent en effet de nouveaux moyens de protection aussi bien que de nouvelles armes. Il s'agit donc, à la fois, de ne pas nous laisser distancer, mais aussi et surtout de nous assurer de l'avance en termes d'initiative technologique. À ce titre, je veux saluer la création de l'Agence de l'innovation de défense, dont nous attendons avec impatience des éléments complémentaires quant à ses moyens et son fonctionnement. La progression des crédits permettra également de répondre à d'autres défis sociétaux et sociaux, notamment par l'investissement de 57 millions d'euros dans le plan Famille. Très attendu par les personnels civils et militaires des armées, celui-ci constitue un levier incontournable de leur fidélisation. Sa mise en place est donc une réelle priorité afin d'assurer un meilleur accompagnement des militaires et de leur famille, notamment sur les questions de mobilité. Concernant le maintien en condition opérationnel- MCO -des matériels terrestres, maritimes et aériens, des efforts importants sont à noter, avec une augmentation de 7 % des crédits par rapport à 2018. Dans une période de fort engagement opérationnel de nos forces armées sur plusieurs théâtres d'opérations, également marquée par la mise en service de nombreux matériels nouveaux, il est primordial que le MCO des équipements soit assuré sans rupture et avec un degré de performance particulièrement élevé, en dépit des contraintes budgétaires et de la complexité des procédures contractuelles. Je tiens cependant à alerter sur la situation de notre marine, qui semble connaître une évolution de ses crédits un peu moins importante que celle des autres forces. Serons-nous à la hauteur avec une augmentation de seulement 6 % pour la préparation des forces navales, alors que cette augmentation est supérieure à 9 % pour les forces aériennes, comme pour les forces terrestres ? À l'heure où la Chine met à la mer l'équivalent de l'ensemble de la flotte française tous les quatre ans, à l'heure où la Russie développe sa capacité de missiles depuis ses navires, il est plus que jamais nécessaire que nous conservions, voire renforcions, nos capacités navales et aéronavales. Elles sont le gage de notre capacité de projection et de notre présence sur tous les théâtres d'intervention au niveau mondial. La conflictualité maritime ne pourra que s'accroître avec le temps et la mondialisation de nos échanges. Ce constat m'amène à rappeler les chiffres concernant le financement des OPEX. Il était en effet prévu une provision de 650 millions d'euros pour les OPEX cette année et 850 millions d'euros en 2019, le reste à financer devant être pris en charge par la solidarité interministérielle. Le général Lecointre, chef d'état-major des armées, avait d'ailleurs rappelé, l'année dernière, que ce complément de solidarité interministérielle était « extrêmement important pour montrer que ce ne sont pas les armées qui décident de leurs engagements ».

Ces OPEX nécessitent, en outre, inéluctablement, un remplacement des matériels les plus anciens par des matériels de pointe. La hausse des crédits répondra, l'année prochaine, aux premiers besoins en la matière.

Derrière ces annonces globalement positives, nous ne pouvons passer sous silence certains points moins satisfaisants du budget dont nous sommes aujourd'hui saisis. Je pense en particulier à l'annulation par le ministère des comptes publics du montant de crédits équivalents à ceux de l'enveloppe interministérielle dédiée aux OPEX. Piochés dans la réserve de précaution sur trois programmes de défense, le 146, « Équipement des forces », le 212, « Soutien de la politique de la défense », et le 144, « Environnement et prospective de la politique de défense », ce sont près de 400 millions d'euros qui disparaissent de la réserve de précaution par un tour de passe-passe budgétaire Pour conclure, madame la ministre, je souhaite rappeler le plein soutien de mon groupe à la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire. Cependant, la coupe claire de crédits opérée par Bercy sur ce budget pour 2019 est inacceptable et incompréhensible. Nos forces ont besoin de ces crédits. Par conséquent, à défaut d'éléments nouveaux, notre groupe s'abstiendra sur le vote des crédits de la mission « Défense ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 11 novembre dernier, au Forum de la paix organisé à la Villette, le Président de la République rappelait notre monde « fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés Comme l'avait souligné le Livre blanc de 2013, puis confirmé La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale en 2017, notre environnement stratégique se durcit. En effet, malgré des décennies de construction d'un droit international, nous ne sommes toujours pas à l'abri des menaces, des menaces qui nous éloignent malheureusement du rêve de Charles Péguy, qui déclarait, à la veille de sa mort, le 5 septembre 1914 : « Je pars, soldat de la République, pour le désarmement général, pour la dernière des guerres. Aujourd'hui, plus de 100 ans après, les défis ont changé de nature, mais, comme hier, ils nous obligent à maintenir et même accentuer l'effort de défense de notre pays. Ces défis, nous les connaissons bien. Il y a celui de la faiblesse des États faillis, qui mobilise nos forces armées, comme c'est, par exemple, le cas actuellement dans la bande sahélo-sahélienne, avec l'opération Barkhane. Il y a celui des postures de puissances de plus en plus affirmées, comme en témoigne la hausse continue des dépenses militaires dans le monde depuis 1999. En 2017, elles ont encore progressé de 1,1 % en valeur. Et je n'oublie pas les menaces de nature contemporaine, en particulier dans les domaines cyber et spatial. À cet égard, nous saluons l'initiative présidentielle lancée au début du mois à l'UNESCO, Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace ». Il y a urgence, car si de nombreux pays, dont la France, ont intégré le cyberespace dans leur doctrine militaire, se pose avec de plus en plus d'acuité la question de la définition de normes communes et de l'application du droit international dans l'espace. Aussi, il faut avancer sur ce dossier sensible. J'en conviens, ce n'est pas facile, comme le laissent entrevoir les discussions en cours à l'ONU, qui se crispent sur les questions de souveraineté et de non-ingérence. Dans ce contexte de menaces protéiformes, les moyens de nos armées doivent être à la hauteur. C'est tout l'enjeu de la nouvelle loi de programmation militaire que le Parlement a adoptée l'été dernier, visant à faire converger le budget de la défense à 2 % du PIB d'ici à 2025. Cela a été souligné par nos collègues rapporteurs, le projet de loi pour 2019 abonde la mission « Défense » de 1,7 milliard d'euros supplémentaires par rapport à 2018, une évolution qui s'inscrit dans la trajectoire fixée par la loi Cependant, alors que celle-ci avait été adoptée à la quasi-unanimité, nous sommes aujourd'hui nombreux à être inquiets, au regard du projet de loi de finances rectificative pour 2018, qui compense le surcoût devenu habituel des OPEX par des annulations de crédits qui sont devenues, elles aussi, habituelles. C'est un mauvais signal, mais j'espère, madame la ministre, que vous nous apporterez des garanties, car il s'agit de garantir la crédibilité de notre défense, et ce à plusieurs égards. Tout d'abord, parce que le respect de la trajectoire budgétaire est bien évidemment une condition de l'efficacité de nos armées. La Revue stratégique l'a constaté : la France a des lacunes capacitaires à réparer. Il n'est donc pas envisageable que les crédits, en particulier, ceux de l'équipement, soient la variable d'ajustement budgétaire, comme cela a déjà été le cas dans le passé. En attendant vos précisions sur la fin de gestion 2018, madame la ministre, pour ce qui concerne les crédits inscrits en 2019 pour l'équipement des forces, on doit reconnaître que l'effort est là, au travers du programme 146 dont les crédits de paiement et d'engagement augmentent significativement. En effet, l'attention portée tant sur les livraisons que sur les commandes devrait permettre de régénérer nos capacités conventionnelles durement éprouvées par la succession J'observe également avec satisfaction l'effort porté sur la Marine qui, on doit bien le dire, a été délaissée par les dernières lois de programmation. Il est important d'inverser la tendance car, d'une part, le défi stratégique en mer s'intensifie, d'autre part, notre pays dispose de la deuxième plus grande zone économique exclusive avec 11 millions de kilomètres carrés. La sincérité budgétaire, nous la devons aussi, et je dirais même « avant tout » aux militaires, hommes et femmes, qui consacrent une grande partie de leur vie au service de la Nation. Nous quittons un cycle mémoriel consacré à la Grande Guerre, et il n'est donc point besoin de rappeler que les militaires, aujourd'hui certes dans d'autres conditions et proportions, risquent néanmoins encore leur vie pour protéger la nôtre. Ce sens du sacrifice, qui est au coeur de leur métier, doit être reconnu. Aussi, je me réjouis de toutes les mesures qui contribuent à améliorer leur quotidien, tant sur le terrain que dans leur vie personnelle. Je pense en particulier aux 57 millions d'euros qui abondent en 2019 le bienvenu « Plan famille 2018-2022 » au sein du programme 212. Enfin, pour terminer, je dirai que c'est également par égard pour nos alliés et nos partenaires que nous devons garantir au mieux une trajectoire budgétaire ascendante pour notre défense. Compte tenu du temps qu'il me reste, je n'évoquerai que nos engagements au sein de l'Union européenne, pour rappeler l'importance de pousser les dossiers de la défense commune pour mieux partager les responsabilités. que vous vous y employez, comme en témoignent vos récentes annonces sur le système de combat aérien futur, le SCAF, pour ne prendre qu'un exemple d'un développement conjoint, en l'occurrence avec l'Allemagne, de capacités futures pour renforcer la défense européenne.

monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de ces présentations et des nombreuses remarques que vous avez bien voulu formuler. J'ai bien noté certaines inquiétudes dans vos propos et je vais y répondre.

Une réponse à des années de réduction de nos moyens, de programmes retardés, de livraisons annulées. C'est une réponse au fossé qui s'est creusé entre nos engagements et les crédits qui étaient accordés pour les remplir. remplir. Ce budget, c'est aussi une ambition pour nos armées. Après une augmentation du budget de 1,8 milliard d'euros en 2018, le PLF 2019 est l'étape suivante pour la remontée en puissance de nos armées, avec 1,7 milliard d'euros supplémentaires. Ce sont donc au total 35,9 milliards d'euros que nous consacrerons à notre défense en 2019, soit 1,82 % de notre PIB.

les attentats de 2015, les armées disposaient en tout et pour tout d'un budget de 32 milliards d'euros. Aujourd'hui, ce sont près de 4 milliards d'euros de plus qui figurent dans ce PLF 2019.

Il s'agit d'actes pour une ambition à « hauteur d'homme », pour le renouvellement de nos équipements, pour l'innovation et pour la préparation des armées aux conflits de demain. Enfin, ce PLF 2019, j'y tiens beaucoup, c'est une responsabilité. C'est l'exigence de finances tenues, une exigence que chaque euro employé soit un euro utile. C'est la nécessité que ces moyens supplémentaires sont bien employés et que nos forces en ressentent au plus tôt les effets. Nous allons donc continuer à moderniser le ministère et je veillerai strictement à la bonne exécution de notre budget. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point dans un instant. Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est un budget de reconquête que je vous présente, d'une reconquête nécessaire pour notre défense, pour nos forces, pour les Français. Car, certains d'entre vous l'ont dit, le contexte international ne s'est pas apaisé. Les menaces restent fortes, violentes, imprévisibles. Nous avons besoin d'affirmer nos alliances et de nous tourner vers l'Europe. Nous avons besoin d'anticiper des conflits sur terre, dans les airs et en mer, mais aussi dans l'espace exo-atmosphérique et le cyberespace. Nous devons faire face, encore et toujours, à la menace terroriste, contre laquelle nos armées combattent à la source. Dans ce contexte, face aux menaces toujours bien présentes, pour répondre aux besoins et aux attentes de nos forces, le PLF 2019 offre des solutions. D'abord pour nos forces, pour leurs familles. Les premiers sacrifices les ont trop longtemps concernés, et cela ne pouvait plus durer. Vous le savez, je tiens particulièrement à mettre l'humain, les civils comme les militaires, les familles, au coeur de notre ministère, au coeur de nos armées, au coeur de notre action. J'ai donc souhaité que le plan Famille entre le plus rapidement possible en vigueur. Je dois dire que je suis très satisfaite de son exécution, qui est le fruit d'un travail tout à fait remarquable mené par nos armées, directions et services. Aujourd'hui, je puis vous dire, comme je m'y étais engagée, que 70 % des mesures du plan ont été lancées, une grande partie a même Quand on parle de wifi qui arrive ou de facilités pour voir son enfant, cela change concrètement la vie. Je ne doute pas que tous ceux qui ont eu l'occasion de rendre visite à nos forces récemment ont pu se rendre compte des améliorations concrètes que tout cela apporte à nos soldats au quotidien. Alors, nous allons continuer et, sans me lancer dans une énumération longue et fastidieuse, je voudrais citer, parmi les mesures du plan Famille pour 2019, un accroissement un accroissement de l'offre de gardes d'enfants, une amélioration de l'accueil des familles, ainsi que des actions de cohésion en garnison ou la pérennisation du dispositif de soutien psychologique aux familles avec l'assistance téléphonique « Écoute Défense ». En 2019, vous l'avez rappelé,

Pour la protection du combattant, ce sont 25 000 gilets pare-balles, des nouveaux treillis, des blindages pour hélicoptères, des moyens de lutte contre les engins explosifs improvisés. Pour la préparation opérationnelle et l'amélioration de la disponibilité du matériel, c'est une augmentation de près de 8 % du budget d'entretien des matériels, porté à 4,2 milliards d'euros en 2019. C'est aussi un effort pour l'amélioration des infrastructures et, en particulier, leur entretien. Comme je vous le disais, et comme vous pouvez le constater, parler de LPM et de ministère à « hauteur d'homme », ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Quand je parle d'actions concrètes, j'en viens assez naturellement au renouvellement de nos équipements, qui est le deuxième axe de la loi de programmation militaire. C''est, comme vous le savez, une nécessité, car nos matériels sont vieillissants pour certains, usés par des engagements intenses dans des milieux particulièrement abrasifs. Alors, il fallait des moyens nouveaux, et il les fallait vite. C'était d'ailleurs le constat que nous avions dressé ensemble voilà quelques mois. En termes de masse budgétaire, ce sont 19,5 milliards de crédits d'équipements qui sont prévus dans le PLF 2019. Je ne vais pas me

qui interviendront pendant l'année 2019, et qui montrent que, non, le renouveau de nos armées ne peut pas attendre, et que, oui, ses effets doivent se faire sentir tout de suite. tout de suite. Pour l'armée de terre, l'année 2019 rime avec l'entrée concrète dans le programme SCORPION, et sera ainsi marquée par la livraison des 89 premiers blindés Griffon. Elle verra aussi la livraison de 8 000 fusils d'assaut HK416, de 50 postes de tir du missile moyenne portée, le MMP, répartis dans 14 régiments, dans 14 régiments, des hélicoptères NH90, très attendus, des parachutes et des véhicules tactiques VT4. Du côté de l'armée de l'air, des équipements indispensables seront livrés, à commencer par le deuxième MRTT, qui viendra s'ajouter à celui qui a été réceptionné le 19 octobre dernier,

d'une frégate multimissions- il y aura donc une FREMM de plus à Brest -, d'un patrouilleur léger et d'un bâtiment multimissions dans les Antilles, ainsi que d'un avion de patrouille maritime rénové Atlantique 2. C'est déjà beaucoup et, pourtant, je n'ai pas tout dit ! Je vous épargne donc les commandes que nous allons lancer, mais elles sont nombreuses, et je compte bien que toutes arrivent dans les temps. Enfin, ce budget fait la part belle aux deux autres axes structurants de la loi de programmation militaire : la préparation aux conflits du futur et l'innovation, avec 758 millions d'euros prévus pour les études en amont, c'est-à-dire une hausse de 5 %. C'est une étape supplémentaire avant d'atteindre le milliard d'euros, dont nous avons parlé ensemble, en 2022. Par ailleurs, les armées disposeront de crédits et d'emplois supplémentaires, les deux tiers étant dédiés aux capacités clés du renseignement, du cyber et du numérique. La force de ce PLF, je voulais le souligner devant vous,

remarques et à vos questions. Il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, tout simplement parce qu'elle est revenue à de nombreuses reprises.

n'ont pas un rapport tout à fait direct avec la réalité. Cette réalité, je vais tenter de vous l'exposer. l'exposer. Tout d'abord, nous avons eu une gestion que je qualifierai de responsable du financement de nos opérations extérieure.

du budget global de notre ministère et que cette annulation s'est imputée sur une réserve que nous avions constituée à cet effet, et que nous avions d'ailleurs qualifiée de « réserve de précaution

je précise qu'aucun gel ni aucun report n'interviendra au moment où nous débuterons la gestion 2019, puisque nous avons obtenu des garanties, avec le dégel, voilà deux semaines, de 272 millions d'euros. Je puis vous confirmer que ces crédits ont effectivement été libérés. Nous respecterons donc le montant voté dans la loi de finances initiale pour 2018 à l'euro près, avec la hausse de 1,8 milliard d'euros du budget des armées, telle qu'elle avait été programmée.

en amorçant une LPM à hauteur d'homme, nécessaire pour nos soldats, nos marins et nos aviateurs, qui s'engagent au quotidien pour la protection de la France et des Français.

Je voudrais enfin insister sur un point, sur lequel nous aurons certainement l'occasion de revenir dans le futur : les décisions de cette année ne font pas les pratiques de demain. Demain, nous entrons dans une nouvelle LPM. Et c'est bien du PLF 2019, le premier PLF de cette nouvelle LPM, dont nous discutons. Aussi, et c'est, je crois, la volonté de tous ici, n'entravons la remontée en puissance de nos armées, n'entravons pas cette augmentation de 1,7 milliard d'euros du budget de la défense pour 2019.

Pour ce qui est des très nombreuses questions que vous avez par ailleurs soulevées, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les orateurs, bien consciente que, dans la minute qu'il me reste, il me sera un tout petit peu difficile de répondre à tout, que ce soit sur les projets d'avenir, le SCAF, la coopération européenne, le programme SCORPION, les réformes structurantes de notre ministère, la nouvelle politique de rémunération des militaires, la réforme des retraites, la poursuite de la réforme du SSA, la mise en oeuvre du prélèvement à la source, la bascule sur, les mesures de fidélisation de nos personnels et et l'évolution du budget de l'ONERA. Je ne peux vous redire qu'une chose : je suis à l'entière disposition de votre commission pour répondre, autant que vous le souhaiterez, lors d'une audition, à la date que vous me fixerez. Pour conclure, permettez-moi de rendre, comme vous, hommage à nos soldats, à nos forces, qui agissent avec courage pour préserver notre souveraineté et nos libertés. Permettez-moi aussi de souligner que nos armées attendent beaucoup de nous tous, de la représentation nationale comme du Gouvernement. Au moment où vous vous apprêtez à vous prononcer sur ce premier budget de la loi de programmation militaire 2019-2025,

Toutefois, plusieurs facteurs sont susceptibles d'entraîner une augmentation substantielle des dépenses de carburant de nos forces armées. En premier lieu, la hausse de la taxation du carburant décidée dans le présent projet de loi, qui devrait, en 2019, faire augmenter le prix du gazole de 7 centimes par rapport à 2018, ce qui revient à une hausse moyenne de 5 %. la hausse du prix du baril de pétrole, qui devrait augmenter d'environ 9,3 % en 2019. Le Gouvernement table sur un prix du pétrole de 73 dollars par baril. Cette prévision ne tient pas compte de la grande volatilité des cours du baril liés à l'évolution du marché, mais aussi aux risques économiques internationaux. Cet amendement vise donc à augmenter de 6 millions d'euros la dotation en carburants opérationnels, afin que ces différents facteurs aient un impact neutre sur le budget de nos forces armées. Cela s'effectuerait par le fléchage de 6 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires

Gouvernement ? Monsieur le sénateur, vous avez raison : les crédits de carburants opérationnels sont essentiels au fonctionnement et à l'activité des armées. Ils font donc l'objet d'un pilotage spécifique par l'état-major des armées. La dotation qui figure dans le projet de loi de finances pour 2019 que j'ai l'honneur de vous présenter s'élève à 458 420 000 euros. Pour dimensionner cette dotation,

dans la loi de finances pour 2018, ainsi qu'un cours de 1,10 euro pour 1 dollar. Pour faire face aux variations du prix du baril, le prix du carburant qui est facturé aux armées par le compte de commerce du service des essences des armées, ou SEA, correspond à un coût moyen unitaire, ce qui permet de lisser le prix d'acquisition sur une longue période. Par ailleurs, le tarif de cession du carburant qui est pratiqué par le SEA prend en compte, outre le cours du pétrole, les coûts d'achat, les coûts de fonctionnement du SEA et l'éventuel recours à un mécanisme de couverture sur les marchés financiers, mécanisme qui fonctionne comme un stabilisateur de prix. Ainsi, l'augmentation du cours du baril de ne se traduit pas, financièrement, par une augmentation immédiate et de mêmes proportions du prix des carburants acquis par les armées.

parce qu'ils sont à 50 % des binationaux, qu'ils sont souvent éloignés des consulats et des ambassades, et que c'est souvent leur seule occasion d'avoir un vrai contact avec les autorités françaises. Supprimer la JDC pour eux, à l'heure où l'on s'apprête à dépenser des millions pour la création d'un service national universel dont ils seront de toute façon exclus, me semblerait une grave faute morale, et stratégique puisque nous avons besoin d'eux comme relais de nos valeurs et comme relais et promoteurs de la francophonie.

que vous avez retiré, considérant avec le Gouvernement qu'il aurait plus sa place dans la mission « Action extérieure de l'État ». C'est la raison pour laquelle je vous suggère, ce soir, d'avoir le même comportement que ce matin

Je vous réponds avec la même conviction que Geneviève Darrieussecq ce matin, en vous assurant combien cette journée est importante pour conforter l'esprit de défense et le lien entre nos armées et la jeunesse.

Par conséquent, je puis vous assurer que nous sommes en discussion avec ce ministère, attachés que nous sommes à la poursuite de l'organisation de cette journée. Je vous serais donc extrêmement reconnaissante de bien vouloir, comme vous l'avez fait ce matin, retirer cet amendement. Nos échanges ne peuvent que conforter la position du ministère des armées pour appuyer, auprès du ministère des affaires étrangères, la poursuite de l'organisation de cette journée.

La séance est levée.